dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. la définition exacte du droit de retrait, droit reconnu par le code du travail dans son article L. 4131-1. C'est précisément ce qu'ont fait valoir les cheminots à la suite de l'accident ferroviaire survenu le 16 octobre, l'avant-veille des congés scolaires. Pour rappel, un autorail TER a percuté un convoi routier, faisant onze blessés. Cet accident grave, et qui aurait pu l'être davantage encore sans l'esprit de responsabilité exemplaire du conducteur, pourtant blessé, a déclenché le droit de retrait de 17 000 cheminots sur les 23 000 conducteurs et contrôleurs, soit plus de 73 % Ces agents ont considéré que les conditions de sécurité n'étaient pas ou plus assurées. Or ni le Gouvernement ni l'entreprise n'ont répondu à leur inquiétude légitime, préférant, par un écran de fumée, relancer un énième débat sur le droit de grève.

La pédagogie de la répétition peut avoir des vertus ; mais elle les perd quand elle consiste à asséner des contre-vérités. En l'occurrence, on ignore l'avis de l'inspection du travail, qui a considéré que le droit de retrait était caractérisé et justifié

que répondez-vous aux inspecteurs du travail, qui recommandent le retour des contrôleurs dans les trains, dans l'attente d'une évaluation complète des risques ? La parole est à M. le Premier ministre. Madame la présidente

À la suite de cet accident, plus de 15 000 conducteurs et personnels de la SNCF ont fait valoir ce que le droit prévoit sous le nom de droit de retrait.

alors que l'accident intervient dans un contexte particulier et sur un type de trains particulier, des conducteurs d'autres matériels à d'autres endroits pourraient considérer que le même problème est susceptible de se poser à eux. Peut-être parce qu'ils rencontrent

pour ne pas respecter les obligations d'information en matière de grève dans les services publics, alors c'est en effet inacceptable- ce sont les mots que j'ai employés -, parce que cela fait peser sur les usagers, sur les familles, sur l'ensemble

Le peuple macédonien l'a fait. Un an plus tard, la France refuse à ce pays l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne. Cette position française illustre un manque de confiance dans la force du projet européen. Elle retire à l'Union européenne une part significative de la crédibilité du processus d'élargissement, donc de son efficacité. ouvre la porte, à nos frontières, à d'autres puissances, qui s'installent parce que nous sommes absents. L'Europe reste un projet, une promesse d'être plus forts ensemble, plus efficacement, solidairement, en affirmant des droits individuels et sociaux. Voilà trente ans, nous avons vu la victoire de peuples européens combattant pour leur liberté et leur indépendance. Cette victoire a permis la réunification de l'Europe. l'Europe. Elle était aussi celle de Charles de Gaulle, de Willy Brandt, de François Mitterrand, qui n'avaient jamais accepté la division, la mise sous tutelle de l'Europe. Nous ne saurions aujourd'hui nous inscrire en rupture de cette vision Monsieur le ministre, l'incertitude sur le Brexit est certes inconfortable, mais une sortie qui gommerait des droits, casserait des règles essentielles à nos libertés, à nos économies, à nos droits sociaux et, vu d'Irlande, à la paix n'est pas acceptable. L'Union européenne peut-elle refuser à Westminster, qui a tant inspiré la tradition parlementaire, un report permettant d'éviter un saut dans l'inconnu ? En le faisant, elle oublierait son rôle essentiel de protection des citoyens. Pourtant, la position française semble aujourd'hui se limiter à l'impatience de tourner la page du Brexit : ce n'est pas convenable. Monsieur le ministre, l'action de la France en Europe vise-t-elle à renforcer une Europe des nations au service exclusif des États membres et de leurs égoïsmes ou une Europe souveraine au service de tous ses citoyens et protégeant leurs droits ?

Nous assumons d'avoir un discours et une stratégie clairs sur le Brexit, parce que nous voulons faire cesser l'incertitude actuelle, extrêmement pénalisante pour des millions de citoyens et de familles : nous voulons les protéger contre cette incertitude qui mine aujourd'hui leurs projets. C'est aussi pour cela que nous avons une position forte en matière d'élargissement, parce que nous voulons que toutes les étapes soient respectées, que les conditions posées voilà dix-huit mois soient respectées. Nous voulons que le processus de négociation soit plus utile, plus transparent, que les populations en bénéficient et stoppent leur émigration massive. Nous voulons une Union européenne qui fonctionne mieux, car, aujourd'hui, à 27 ou à 28, nos décisions sont

Madame la secrétaire d'État, si l'action de la France était conforme à ses paroles, crédible et comprise, nous n'aurions probablement pas eu à subir le camouflet du refus de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne

Droit de grève ou droit de retrait, tous les moyens sont bons ! Nous avions connu, en 2018, la grève perlée, la grève capillotractée des jusqu'au-boutistes. Nouvel épisode, même saga ; nouvelle recette, même tambouille. Mercredi dernier, un accident à un passage à niveau dans les Ardennes a fait onze blessés, dont le mécanicien, seul agent SNCF à bord. Cet accident a été particulièrement violent, et on ne peut remettre en question l'émotion légitime qu'il a suscitée. Il fait l'objet de plusieurs enquêtes : il faudra notamment déterminer pourquoi le système radio sol-train n'a pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le droit de retrait n'a pas été limité à certains matériels identifiés comme éventuellement porteurs de failles de sécurité- certains systèmes étaient déjà utilisés dans les années 1970. Il n'a pas été limité non plus, madame Assassi, aux lignes sans contrôleur les TGV et les Intercités ont aussi été touchés. Ce droit de retrait a été étendu à tout le territoire national. La spontanéité de l'émotion a manifestement été exploitée et récupérée. Les syndicats espéraient peut-être la sympathie des usagers ? Savant calcul ! Les centaines de milliers de voyageurs bloqués lors d'un week-end de départs en vacances sont évidemment excédés. excédés. S'agissait-il plutôt d'un test pour le 5 décembre ? Vous savez, ce jour où les syndicats protesteront contre une réforme dont le contenu n'est pas encore connu ! La confusion des demandes mêlée à une disproportion totale démontre l'abus du droit de retrait. D'ailleurs, le danger grave et imminent a, semble-t-il, disparu, puisque le travail a repris, sans qu'on sache ce qui a changé depuis mercredi dernier. C'est le caractère inique de ce mouvement ! Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que ces dérives inacceptables seront sanctionnées, afin que le droit de retrait ne devienne pas la façon commode de détourner la grève ?

comme le week-end dernier, pour partir en vacances. Quand on dit défendre le service public, on doit penser d'abord aux usagers ! La grève est un droit, que personne ne remet en question, mais il existe des procédures permettant aux salariés de faire valoir leurs revendications et d'exercer leurs droits en minimisant la gêne pour les usagers. Clairement, ces procédures n'ont pas été respectées. Le trafic est aujourd'hui revenu à la normale, sauf dans les Ardennes et les départements voisins. C'était notre objectif principal. La SNCF a annoncé des mesures exceptionnelles pour indemniser les voyageurs

est la première priorité pour tout le monde, pas seulement pour les syndicats. C'est le sens des enquêtes qui ont été lancées au sein de la SNCF et de l'enquête que Jean-Baptiste Djebbari et moi-même avons demandée au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. C'est le sens aussi des engagements qui ont été pris immédiatement par

Républicains. Monsieur le ministre de l'intérieur, il y a dix-huit jours, la France était en état de choc à la suite de la tuerie de quatre membres de la préfecture de police de Paris par un fonctionnaire radicalisé. Il a fallu plusieurs jours- non sans cafouillages et avec des pudeurs sémantiques-, plusieurs jours de balbutiements politiques, malgré la réactivité des enquêteurs, pour admettre que l'assassinat reposait sur des motifs religieux. Certes, deux missions ont été annoncées à juste titre par le Premier ministre pour détecter les agents radicalisés dans les services antiterroristes. L'une de ces missions est relative à la fameuse direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, qui, dès 2015, aurait dû s'apercevoir du changement d'apparence et de comportement de ce fonctionnaire. La réorganisation ou le rattachement de la DRPP s'impose. Près de trois semaines après cette tuerie, rien n'a été fait. Les Français demandent des décisions immédiates, au moment où le Gouvernement a reconnu cette sécession insidieuse qui menace la société. Les dérives communautaires de certains employés de service public exposés sont alarmantes. Par la bien-pensance des élites, des signes évidents de radicalisation dans ces services sont tus. C'est même le mot radicalisation qui fait peur : on n'ose pas désigner l'ennemi, alors que nous sommes en lutte contre l'islamisme politique. Comme l'a dit Bruno Retailleau, le communautarisme prépare le terreau des vocations djihadistes de demain. À chaque problème, l'exécutif tempère. Nous sommes devenus coutumiers de cette indécision permanente, là comme dans bien des domaines. Monsieur le ministre Castaner,

Immédiatement, le Premier ministre a saisi l'inspection des services du renseignement de deux missions. La première vise à comprendre comment le signalement concernant M. Harpon n'est pas remonté dans la hiérarchie et n'a pas été traité comme il aurait

Quel est ce dispositif dans les services de police ? Il est très simple : c'est au chef de service de police qu'il revient de procéder aux signalements puis de les faire remonter à l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, qui, en liaison avec certains services de renseignement, dont la direction générale de la sécurité intérieure,

pour le groupe Union Centriste. Madame la ministre, le 89 congrès de l'Assemblée des départements de France, qui a eu lieu à Bourges la semaine dernière, s'est soldé par un échec. Les discussions avec le Gouvernement ont achoppé sur la question de l'avenir de la fiscalité départementale. Réforme après réforme, les élus départementaux ont le sentiment que leur circonscription s'apparente, non plus à une collectivité décentralisée de plein exercice, mais à un échelon déconcentré de l'État. Le transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale, inscrit par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2020, traduit ce lent processus de recentralisation financière amorcé voilà bientôt dix ans par la suppression de la taxe professionnelle, et prolongé depuis par la suppression d'une partie de la CVAE dans le cadre de la loi NOTRe. En leur retirant la dernière imposition sur laquelle ils avaient encore un pouvoir de taux, le Gouvernement s'apprête à réduire comme une peau de chagrin l'autonomie fiscale des départements. Cela est d'autant plus vrai que vous semblez écarter tout déplafonnement des droits de mutation à titre onéreux. L'attribution d'une fraction compensatoire de la TVA offrira certes une ressource dynamique, mais elle sera nécessairement plus sensible aux variations de la conjoncture économique. Elle pourrait en outre être affectée par des décisions qui, étant prises au niveau national, échapperaient à la responsabilité des élus départementaux. Alors que les départements engagent chaque année pour le compte de l'État 11 milliards d'euros de dépenses sociales, comment pouvez-vous, madame la ministre, garantir aux conseils départementaux une évolution des transferts fiscaux qui soit à la hauteur des charges qu'ils assument pour le compte de la Nation ? La parole

le système est plus équitable. Il faut insister sur ce point : riche ou pauvre, quelle que soit la dynamique foncière, chaque département verra progresser de la même manière ses ressources chaque année.

Premièrement, la fraction de TVA ne prendra malheureusement pas en compte l'évolution démographique et l'effort de construction de chaque département. Deuxièmement, il serait légitime qu'en cas de baisse du produit de la TVA à l'échelle nationale

dont 1 milliard pour la France. Cela fait suite à une décision de l'OMC relative au financement des développements d'Airbus. Je ferai trois remarques.

Enfin, à ma connaissance, le gouvernement fédéral américain déverse des centaines de milliards de dollars dans l'industrie aéronautique américaine sous prétexte de contrats d'étude et de recherche.

Sans doute aurons-nous à prendre des mesures de sauvegarde ou de compensation pour les exportateurs français. Peut-être pourrez-vous nous en dire un mot, madame la secrétaire d'État ? L'OMC devrait donner la possibilité à l'Europe d'imposer des sanctions en

L'Union européenne serait fondée à imposer des droits de douane contre les États-Unis dans le contentieux parallèle contre Boeing, mais le calendrier n'est pas très favorable puisque nous attendons la confirmation

de ces contentieux. L'escalade des tensions avec un allié et un partenaire ne nous semble pas souhaitable, car elle aurait un impact encore plus négatif sur nos économies, notre commerce et notre industrie aéronautique. Nous continuons donc à proposer aux États-Unis de dialoguer.

Nous regrettons que les États-Unis aient jusqu'ici refusé d'engager les discussions vers un compromis. J'appelle très solennellement devant vous l'administration américaine à entamer des négociations le plus vite possible, sans quoi nous prendrons des mesures de rétorsion.

La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le Premier ministre, l'organe de règlement des différends de l'OMC a confirmé la semaine dernière qu'il autorisait les États-Unis à augmenter les taxes sur les biens et les services européens dans le cadre du dossier des subventions Airbus. Le président Trump a choisi de réserver un traitement de faveur au deuxième poste, excédentaire de 11,7 milliards d'euros, de notre balance commerciale française : le vin.

La viticulture française est aujourd'hui la victime collatérale d'un conflit industriel qui ne la concerne pas. C'est une nouvelle épreuve pour une filière entrée dans une forte zone de turbulences. À l'étranger, nos marchés sont moroses instabilité politique à Hong Kong, obligeant à l'annulation du Wine Festival ; interminable Brexit ; écroulement du marché chinois sur lequel, il y a cinq ans, la viticulture faisait déjà les frais d'un conflit avec l'Union européenne sur les panneaux photovoltaïques ; contexte national en berne, également. Attaquée de toutes parts sur ses propres terres par l'urbanisation rampante, par la pression sociétale sur l'environnement et la traçabilité des produits, mais aussi par la raréfaction de la main-d'oeuvre et les problématiques de transmission, le modèle viticole français est sérieusement ébranlé. Le « viti-bashing » fait son oeuvre et sape le moral des vignerons. La filière viticole fait pourtant tant d'efforts ... Malgré les déchaînements climatiques, elle concourt largement à ce que la France soit, pour la troisième année consécutive, considérée comme ayant l'alimentation la plus durable du monde. Que faire, monsieur le Premier ministre, pour le vin, qui occupe une place si particulière dans la culture française ainsi que dans notre économie, puisque la filière représente plus de 500 000 emplois directs et indirects ? Les élus du vin et des terroirs, regroupés au sein d'une association dont je suis la coprésidente, vous ont proposé il y a quelques semaines l'organisation en urgence d'un Grenelle de la viticulture. Allez-vous y répondre par l'affirmative ? La parole

les solutions de compromis, mais nous ne sommes pas totalement assurés qu'elles arrivent immédiatement. Aussi avons-nous essayé de mobiliser à la fois la Commission européenne et des positions françaises. Lors du conseil des ministres de l'agriculture du 14 octobre dernier, je suis intervenu au nom de l'Italie, de l'Espagne et de la France pour solliciter

pour lui demander que la Commission finance la mise en oeuvre rapide des programmes de promotion- c'est absolument indispensable ; que des garanties soient apportées aux opérateurs mettant en oeuvre ces mêmes mesures, parce qu'aujourd'hui les opérateurs sont sur la brèche

Ce pays, miné par le développement du terrorisme islamique, est au bord de l'effondrement. Un tiers de son territoire est déjà aux mains des djihadistes. Alors que, selon l'ONU, on comptait fin août 290 000 déplacés, ils seront probablement 500 000 à la fin de l'année ; 3 000 écoles sont déjà fermées, de même que tous les hôpitaux et dispensaires des zones concernées. Le pire est que l'influence des terroristes ne cesse de grandir. Désormais, ce sont des attaques quasi quotidiennes qui frappent le pays, avec leur cortège de pertes humaines, militaires et civiles. L'armée nationale est malheureusement impuissante à endiguer cette progression. Le risque est de voir le scénario malien se rejouer dans ce pays. Cela est d'autant plus grave que le Burkina Faso n'est pas n'importe quel pays : il est assurément un verrou stratégique pour bloquer l'expansion du terrorisme vers les pays du golfe de Guinée, tels que le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana qui s'inquiètent à juste titre. Les pays de la Cédéao ont d'ailleurs solennellement tiré la sonnette d'alarme lors d'un sommet extraordinaire mi-septembre à Ouagadougou. Monsieur le Premier ministre, mes questions à cet égard sont simples. Tout d'abord, cinq ans après le succès de l'opération Serval, qui avait permis d'empêcher le renversement de l'État au Mali, de la gravité de la situation au Burkina Faso, que compte entreprendre la France ? Ensuite, le Président de la République a annoncé à la fin de l'été « un nouveau partenariat pour la sécurité et la stabilité au Sahel », », qui peut assurément concerner des pays européens, mais également la Cédéao, laquelle s'est notamment engagée à financer une nouvelle force régionale à côté du G5 Sahel : pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? Enfin,

les victimes civiles et militaires se multiplient également puisque, le week-end dernier encore, quatre militaires et un policier ont été tués. Vous décrivez aussi une détérioration de la situation humanitaire. C'est une réalité : on dénombre 250 000 déplacés et, peut-être, 1,2 million de

Le fait que la quasi-totalité des présidentes et présidents des départements de France ait quitté la salle lors de leur congrès annuel, alors que la ministre représentant le Gouvernement s'exprimait, est pour le moins inhabituel et lourd de sens. Ces élus, dans leur diversité politique, ont ainsi voulu dénoncer la mise sous tutelle des budgets départementaux, engagée avec le pacte de Cahors fin 2017 et confirmée dans le projet Ils s'inquiètent à bon droit de la fin de leur autonomie fiscale avec le transfert de la taxe foncière aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Ils ne se satisfont pas de l'octroi d'une part de TVA en compensation de cette perte, et ce pour trois raisons. Vendu comme dynamique par le Gouvernement, cet impôt est de fait très aléatoire. De plus, son rendement s'inverse mécaniquement en période de crise, alors même que toute crise engendre plus de précarité et donc plus de dépenses de solidarité versées par les départements.

Enfin, ils dénoncent la remise en cause inacceptable de l'histoire et des principes de la décentralisation la mise à mal de leur autonomie financière et fiscale. Quelle suite le Gouvernement entend-il réserver à leurs légitimes inquiétudes ?

plutôt que de maltraiter les départements, de travailler avec eux, à leurs côtés, chacun à sa place, chacun dans son rôle, pour plus de cohésion sociale et territoriale

ce sont des contraintes supplémentaires, des charges supplémentaires, 80 intrusions dans des élevages pour démontrer la maltraitance des animaux ! En revanche, jamais on n'a diffusé de vidéo montrant un agriculteur pleurer devant un animal qui venait de périr.

je partage votre inquiétude. Je souhaite vous dire que le Gouvernement est tout entier derrière les agriculteurs lorsque ceux-ci sont montrés du doigt,

unanime du monde agricole, des industries agroalimentaires, des entreprises de transformation, des coopératives et des responsables politiques de changer la façon de faire. que la première chose à changer, c'était le prix payé aux agriculteurs. Il est absolument inacceptable qu'un agriculteur vende son lait et sa viande au-dessous du prix de revient, de ce que cela lui

Ma question s'adresse à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur la décision de supprimer, à compter du 31 décembre 2019, le prêt à taux zéro « logement neuf » pour les habitants des zones B2 et C, c'est-à-dire dans les villes moyennes et les secteurs ruraux. Selon le Gouvernement, cette non-reconduction répondrait à un double objectif : d'une part, revitaliser les centres-bourgs anciens, et, d'autre part, lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. En effet, le prêt à taux zéro, serait maintenu dans ces deux zones pour l'achat dans l'ancien jusqu'en 2021. Pourtant, la fin de ce dispositif risque de mettre un coup d'arrêt à l'accession à la propriété pour les jeunes familles et, par conséquent, de pénaliser le secteur du bâtiment. En outre, cette disparition irait à l'encontre des objectifs du Président de la République, qui a fait de la réduction des inégalités territoriales et du développement harmonieux et équilibré des territoires l'une des priorités de son action, la mise en place de l'agenda rural que vous portez, madame la ministre, devant concrétiser et ancrer dans la durée les actions du Gouvernement en faveur des ruralités. Réserver ce PTZ dans le neuf aux grandes métropoles, à une partie de la Côte d'Azur, ou encore au seul périmètre aggloméré de l'Île-de-France, soit les zones serait un très mauvais signal pour débuter l'agenda rural. Je vous demande donc de bien vouloir réexaminer ce dossier et de maintenir le dispositif du prêt à taux zéro dans les zones B2 et C.

de recentrer progressivement le PTZ dans le neuf sur les zones les plus tendues, là où le besoin en logements neufs est le plus fort pour nos concitoyens. Afin de donner de la visibilité aux professionnels, nous avons toutefois fait le choix de reconduire le dispositif pendant deux ans dans les zones B2 et C, avec une quotité de 20 %. Pour ce qui concerne le PTZ dans l'ancien, nous l'avons recentré sur les zones les moins tendues, car c'est dans ces territoires que les besoins en termes de rénovation sont les plus forts.

cela évite de consommer de l'espace et de l'artificialiser et, enfin, parce que cela permet de faire revenir des habitants dans les centralités des villes moyennes et des petites villes. Tout cela va dans le sens des programmes « Action coeur de ville » et « Petites villes de demain » que nous allons lancer notamment dans le cadre de l'Agence prendre une nouvelle décision sur le PTZ dans le neuf, le Gouvernement a donc souhaité s'accorder le temps de la réflexion et disposer d'analyses précises. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé un rapport d'évaluation qui sera remis prochainement et qui permettra d'éclairer le débat parlementaire. Sur le fondement de ce travail et des orientations fixées, notamment dans l'agenda rural, comme vous l'avez rappelé monsieur le sénateur, de nouvelles pistes pourront être explorées et mises en oeuvre. Je pense en particulier à la prolongation du PTZ pour de gros travaux assimilés à du neuf. La parole

À l'automne, sont organisées dans les territoires alpins et pyrénéens les grandes foires agricoles, celles où éleveurs, maquignons et bergers se retrouvent le temps d'une journée pour partager les dernières anecdotes de la saison d'estive et vendre leurs bêtes. des agneaux, des veaux qui n'ont pas encore connu les étables : des bêtes élevées en plein air, avec soin et, j'ose le dire, avec amour ! Cette année pourtant, à la traditionnelle foire aux tardons du Haut-Champsaur, il était impossible d'acheter des brebis. Malgré la qualité des produits locaux, malgré le soleil et les couleurs d'automne, le temps n'était pas à la fête. D'ailleurs, de nombreux maires venus des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, de Vaucluse et des Alpes-Maritimes s'étaient rendus jusqu'à Champoléon pour exprimer leur soutien aux éleveurs, et interpeller les pouvoirs publics sur une réalité qui n'est plus tenable. En effet, dans certains alpages comme ceux qui sont situés au coeur du parc national des Écrins, il est impossible d'appliquer les mesures de protection du plan national d'actions sur le loup et les activités d'élevage.

La question n'est pas de savoir qui du ministre de la transition écologique et solidaire ou du ministre de l'agriculture et de l'alimentation aura le dernier mot. Non, monsieur le Premier ministre, la question est de savoir si la France veut ou non maintenir la tradition du pastoralisme et la vie qui va avec ! La parole est à M. le ministre de l'agriculture

ce n'est pas suffisant ! Il est temps que le Gouvernement prenne ses responsabilités et assume ses choix. Il est temps que les paroles soient en adéquation avec les actes. Il est temps que le Gouvernement explique aux consommateurs qu'il n'est pas favorable à l'élevage extensif, préférant abandonner la montagne au loup et à l'ours.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire. Madame la ministre, comme vous l'avez annoncé en juillet dernier et conformément aux préconisations de la mission d'information sur le désenclavement des territoires par le transport aérien, dont j'ai été la rapporteure, les vols vers les territoires ultramarins et la Corse, ainsi que les lignes d'aménagement du territoire sous obligation de service public, seront exemptés de la hausse de la taxe de solidarité prévue dans le projet Mais un amendement déposé par le Gouvernement et adopté à l'Assemblée nationale tend à subordonner cette exonération à une décision de la Commission européenne, permettant de considérer ce dispositif législatif comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

du tout. Vous le savez, madame la ministre, ces vols sont indispensables à l'aménagement du territoire et une hausse de la taxation mettrait en danger leur équilibre économique, extrêmement fragile.

C'est une réponse apportée à nombre de nos concitoyens, qui nous ont expliqué ne pas comprendre pourquoi ils payaient une fiscalité carbone sur leur carburant tandis que d'autres Français n'en paient pas sur le transport aérien.

les deux tiers en seront payés par des compagnies étrangères. Je rappelle qu'une telle contribution existe déjà dans de nombreux pays et que nous sommes le seul à la moduler

Je vous remercie, madame la ministre, pour ces propos rassurants. Vous savez combien ces lignes d'aménagement du territoire sont importantes pour nos territoires isolés,

Quelques mois plus tard, alors que deux compagnies françaises- Aigle Azur et XL Airways -annoncent leur faillite, laissant sur le carreau plus de 1 700 salariés, le Gouvernement propose une hausse de la taxe de solidarité d'environ 200 millions d'euros sur les billets d'avion. Une disposition fiscale qui n'est, en réalité, qu'une variable d'ajustement budgétaire. Peut-être, madame la ministre, y a-t-il entre nous un malentendu sur la définition donnée à la notion de compétitivité ou peut-être la politique du Gouvernement manque-t-elle de cohérence, voire de vision stratégique

Mes questions sont donc simples. Avez-vous abandonné l'objectif de redresser la situation du transport aérien français ? Avez-vous également abandonné vos ambitions environnementales, en préférant utiliser la taxation de l'aérien comme une variable d'ajustement budgétaire plutôt que comme un véritable levier d'accompagnement du secteur, dans la recherche et développement et, plus particulièrement, pour la structuration d'une filière de bio-carburant, comme nos compagnies aériennes

le carburant de leur voiture, alors que le kérosène en est exempté. Je pourrais ajouter qu'ils ne paient pas non plus de TVA sur les vols intérieurs, contrairement aux trains internationaux. C'est dans ce contexte et, en effet, pour financer une politique

ou au Royaume-Uni qu'en France. Je rappelle au passage que l'Allemagne vient de décider d'augmenter la taxe sur ses propres billets de 74 %.

continuer à faire de ce mode de transport un levier de puissance, pour préparer notre industrie à l'avion de demain. L'État se doit d'accompagner la mutation technologique et environnementale du secteur aérien, en soutenant massivement la recherche et le développement, la structuration d'une filière de bio-carburant. C'est cela une vraie politique éco-responsable ! N'oublions jamais que les compagnies aériennes sont la marque d'une grande nation. Vecteurs majeurs du désenclavement du territoire, de notre lien avec le monde, elles sont essentielles à notre rayonnement

11 blessés. Malgré son état de choc et ses blessures, le conducteur a aidé les passagers blessés, dont plusieurs ont été hospitalisés. Avec sang-froid, et seul, il a évité de justesse un sur-accident qui aurait pu s'avérer dramatique pour les 80 passagers. Il a effectivement longé les voies sur plus d'un kilomètre pour avertir le train suivant. Le drame a donc été évité grâce à la conscience professionnelle de ce conducteur attaché à son métier, qui a d'ailleurs tenu à rester discret. Malheureusement, cet accident met en lumière

La disparition des contrôleurs et des moyens humains n'est pas la bonne solution. Nous aimerions donc connaître votre position sur ce point. Quels moyens sont mis en place pour lutter contre la fraude dans les trains dépourvus de contrôleur ? Cet accident rappelle également la dangerosité des passages à niveau.

pour son très grand professionnalisme. Il a eu les bons réflexes pour assurer la sécurité des voyageurs. La sécurité est aussi notre priorité absolue, et c'est le sens des enquêtes qui ont été lancées, aussi bien au sein de l'entreprise que par mon ministère, le

à Limoges. Dans ces conditions, on peut se dire que l'on était bien loin du droit de retrait ! Nous sommes tous attachés à la sécurité ferroviaire, au respect du droit de grève, comme nous sommes tous attachés au service public. Cela signifie, aussi, penser aux usagers

la demande du groupe socialiste et républicain, la discussion de la proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXI siècle, présentée par

avec détermination les orientations fiscales et budgétaires du Gouvernement. Cette proposition de loi sur les successions et les donations s'inscrit dans cette perspective. Pris dans sa version initiale- ce ne sera plus vraiment le cas à la fin de notre discussion,

présenter nos positions à l'issue de l'examen en commission de notre texte, pour me concentrer, en tant qu'auteur, sur l'esprit général de notre proposition de réforme de la fiscalité des successions et donations.

Les études récentes, dont celle, très actuelle, de Thomas Piketty, convergent à montrer que le creusement constaté est d'abord lié aux inégalités de patrimoine, plus qu'aux inégalités de revenu, sans pour autant les oublier. Autrement dit, le fautif n'est pas tant notre système social redistributif que la que la reproduction patrimoniale systématique et amplifiée. C'est contre ce phénomène dit « des héritiers », trop bien connu et trop souvent laissé de côté, que nous souhaitons nous engager aujourd'hui avec cette proposition de loi. Cette dernière repose sur deux principes : favoriser une redistribution intragénérationnelle, par des mesures visant à taxer davantage les gros patrimoines, et une redistribution intergénérationnelle, par des mesures favorisant les successions et donations familiales. Si, pour nous, ces deux préoccupations doivent être liées pour une réforme globale et efficace- d'où notre texte -, nous avons bien compris la difficulté de les faire valider toutes les deux par notre assemblée. Je veux donc revenir plus en détail sur ces deux principes, plus spécifiquement sur le deuxième, sur lequel la commission s'est accordée, ce dont je me réjouis. S'agissant de la redistribution intragénérationnelle, notre objectif notre objectif assumé est de taxer davantage les plus hauts patrimoines de notre pays lorsqu'ils sont transmis. C'est dans cette perspective que nous proposons une augmentation de la progressivité des droits de mutation et l'élargissement de l'assiette, avec l'intégration des assurances vie et la suppression de quelques niches patrimoniales. Ces mesures, mes chers collègues, sont nécessaires pour mieux taxer les forts patrimoines lors des successions, qui sont la cause directe de l'accroissement des inégalités sociales et économiques, comme précédemment expliqué. Ce sont ces mesures qui visent le plus directement à mieux redistribuer entre nos concitoyens. Nous avons d'ailleurs également proposé la prise en compte des héritages antérieurs dans le calcul de ces droits, pour mieux contrer ceux qui contournent le système actuel : l'optimisation patrimoniale et successorale est un des grands travers de notre système actuel de succession. C'est aussi par réalisme, et parce que nous ne croyons pas aux solutions confiscatoires, que nous avons proposé un système équilibré : davantage taxer les gros patrimoines, encore une fois par l'élargissement de l'assiette et une plus grande progressivité, mais aussi

Notre article d'augmentation de l'abattement général a d'ailleurs pour sens de prendre en compte l'explosion du prix de l'immobilier actuel, notamment en zone urbaine. Telle est notre volonté générale sur le plan de la redistribution intragénérationnelle, qui est, pour nous, une priorité pour lutter contre les inégalités. Le rapporteur a proposé un certain nombre de suppressions et modifications, sans surprise compte tenu du clivage droite-gauche existant dans notre Haute Assemblée et toujours aussi vivace dans

Ce deuxième pilier de notre proposition de loi est fondamental si nous voulons, demain, permettre une circulation plus aisée, plus importante des patrimoines, notamment des petits patrimoines.

Ce recul progressif de l'âge d'héritage est naturellement le résultat de l'allongement de la durée de vie. Mais il a de réelles conséquences sur la mobilité des patrimoines et l'utilisation des

cette disposition permettrait aux grands-parents de choisir comment organiser leur succession, ce qui est impossible aujourd'hui compte tenu du trop faible abattement prévu en cas de saut de génération. On permettrait ainsi aux petits patrimoines d'aider leurs petits enfants âgés de 20 à 30 ans pour construire leur vie. Cette simple mesure de solidarité intergénérationnelle à destination des jeunes serait, à la fois, un signal fort pour l'insertion des jeunes et pour la circulation patrimoniale. Cette mesure ferait date car elle serait en car elle serait en faveur de la jeunesse de ce pays, qui est en attente d'un message en sa direction, désespère de voir une réelle reconnaissance, aspire à construire la société

Enfin, mes chers collègues, je veux revenir sur le lien entre nos deux objectifs. Si nous proposons aujourd'hui ce mécanisme intergénérationnel, c'est pour aider les grands-parents ayant péniblement cumulé un bien dans leur vie à soutenir leurs petits-enfants. Mais nous ne souhaitons pas que ce dispositif soit utilisé, comme tout le reste du dispositif de succession et donation, par certaines plus grosses fortunes pour léguer sans être taxées. C'est pourquoi je veux insister sur les autres articles de ce texte, qui, demain, pourraient être des garde-fous pour les héritages des enfants ou des petits enfants. Par ce texte, nous espérons que le Gouvernement comprendra qu'un autre chemin est possible que le sien, qui, pour l'instant, a privilégié les plus aisés de nos concitoyens. Un chemin qui permette d'aider les jeunes, tout en faisant contribuer les gros patrimoines. Un chemin qui redistribue, tout en préservant les classes moyennes. Un chemin qui favorise la lutte contre les inégalités, que le système actuel laisse manifestement perdurer.

Une fiscalité qui tienne compte de la réalité de notre pays, de son évolution démographique, des changements des structures familiales et des écarts de richesses. C'est tout l'esprit de cette proposition de loi. La parole est à M. le rapporteur.

je tiens d'abord, une nouvelle fois, à saluer le travail effectué par les auteurs de la proposition de loi, en premier lieu MM. Thierry Carcenac et Patrick Kanner, et ce en dépit de nos divergences de vues. Les échanges passionnés que nous avons eus en commission la semaine dernière traduisent clairement la nécessité de reposer la question du juste niveau d'imposition de la transmission du patrimoine, qui n'a plus été abordée depuis 2012. Il s'agit pourtant d'un sujet majeur, tant pour les finances publiques que pour nos concitoyens. Du point de vue budgétaire, les droits de mutation à titre gratuit, les DMTG, ont effectivement rapporté l'an passé 16,2 milliards d'euros, dont 2,7 milliards d'euros au titre des seules donations. Deux constats relatifs au poids des DMTG peuvent être dressés. D'une part, leur rendement apparaît très dynamique, puisque leur poids dans la richesse nationale a triplé depuis 1965. D'autre part, les comparaisons internationales suggèrent que la France « surtaxe » les successions et donations. Notre pays arrive ainsi en deuxième position, juste derrière la Belgique, lorsque l'on classe les pays selon le rendement des droits de succession et de donation. Du point de vue du consentement à l'impôt, il n'est par ailleurs pas inutile de rappeler que les Français font preuve d'une grande défiance à l'égard de cette forme de taxation. Ainsi, une récente étude réalisée par France Stratégie révèle que « la grande majorité des personnes interrogées- 87 % -se prononce en faveur d'une diminution de la taxation des héritages », y compris ceux qui estiment avoir peu de chances d'hériter un jour. Enfin, le débat relatif à la fiscalité des donations et des successions s'inscrit dans un contexte social renouvelé, dans la mesure où l'âge moyen auquel on hérite a fortement reculé, cela a été rappelé, pour atteindre désormais 50 ans. S'il s'agit d'une évolution heureuse, cela a pour conséquence que l'héritage intervient trop tardivement pour aider à démarrer dans la vie. C'est à l'aune de ces constats que la commission des finances a examiné la proposition de loi mercredi 16 octobre. Sur le plan de la procédure, il peut être souligné que le texte a fait l'objet d'une législation en commission- ou LEC - partielle pour les articles 3, 4, 5, 9 et 10, à la demande du groupe socialiste et républicain. Jamais une proposition de loi issue de l'opposition n'avait fait l'objet d'une LEC partielle. Dès lors, la question de l'articulation de cette procédure avec la pratique du s'est posée. posée. Avec l'accord du groupe socialiste et républicain, la commission des finances a finalement amendé l'ensemble des articles dès le stade de l'examen en commission, afin d'éviter un rejet global du texte, qui aurait abouti à un retour à la procédure normale sur l'ensemble des articles. Sur le fond, la commission des finances a adopté une « grille d'analyse » pouvant être déclinée en trois axes. Premièrement, toutes les initiatives augmentant les droits de mutation à titre gratuit ont été écartées. Compte tenu du poids élevé des DMTG en France et de leur impopularité, il ne nous a pas semblé souhaitable de renforcer la fiscalité des successions et donations, et ce y compris en rabotant les niches fiscales, telles que le « pacte Dutreil », qui ne sont que le corollaire indispensable au haut niveau global de de taxation. Pour cette raison, la commission des finances a supprimé les articles 4, 5, 7, 8 et 9. Ces articles visaient notamment à revenir sur la fiscalité dérogatoire de la transmission des sommes issues des contrats d'assurance vie, ou encore à supprimer des exonérations de DMTG sur les bois et forêts. Deuxièmement, les propositions trop coûteuses du point de vue des finances publiques ont également été écartées. Dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances, la commission a considéré que nous ne pouvions pas reprocher au Gouvernement de ne faire aucun effort de redressement des comptes publics en adoptant, dans le même temps, des amendements dont le coût se chiffrerait en milliards d'euros. Pour cette raison, la commission a modifié les articles 1 et 6 afin d'introduire des dispositifs plus ciblés- nous y reviendrons. Troisièmement, l'objectif d'encourager la circulation anticipée du capital vers les jeunes générations a constitué la priorité de la commission des finances. Dans un contexte de forte hausse des prix des logements et d'allongement de la durée des études, il paraît évident que la solidarité familiale entre les générations doit jouer un rôle décisif pour aider les jeunes à financer leurs études et à se constituer un premier apport pour devenir propriétaires. En conséquence, nous avons souhaité encourager fortement les donations vers les petits-enfants. La commission des finances a ainsi adopté des modifications aux articles 1 et 2 visant à renforcer significativement l'abattement sur les donations aux petits-enfants et à diminuer le délai de rappel fiscal pour les moins de 40 ans, dans le même esprit que les auteurs de la proposition de loi. Au total, c'est donc une proposition de loi équilibrée et recentrée sur l'objectif de venir en aide aux plus jeunes qui émerge des travaux de la commission des finances ! La parole

je le dis d'emblée, comme je l'ai dit en commission la semaine dernière : le Gouvernement est attaché à l'équilibre qui caractérise aujourd'hui la taxation des donations et des transmissions. Depuis leur instauration, au lendemain de la Révolution française, les droits sur les successions et les donations ont été conçus comme un instrument de redistribution afin d'éviter la concentration du patrimoine. patrimoine. Devenus progressifs à compter de 1901, les droits de mutation à titre gratuit, ou DMTG, sont construits sur la prise en compte du couple défunt-héritier ou donateur-donataire, en favorisant les liens de parenté les plus proches. Les droits de succession et de donations relèvent d'un barème progressif, mais aussi des divers abattements ou exonérations favorables aux transmissions familiales. Du fait de la limitation des donations antérieures à quinze ans, ces dispositions permettent une transmission préparée et anticipée pour réduire les droits dus en faisant jouer, tous les quinze ans, le même abattement. même abattement. Dès lors, le régime des donations et successions aboutit déjà à une franchise d'impôt pour la grande majorité des transmissions en ligne directe. En effet, ces dernières bénéficient d'un abattement de 100 000 euros : ce n'est qu'au-delà de cet abattement que s'applique le barème progressif d'imposition selon le montant du patrimoine transmis par part. Cet abattement est lui aussi valable sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants. Ainsi, pour un couple avec deux enfants, il est aujourd'hui possible d'effectuer une donation de 400 000 euros sans payer de droits, soit 100 000 euros pour chacun des parents, et pour chacun des deux enfants.

Dans la version initiale de ce texte, rien n'aurait empêché à chacun des deux grands-parents de transmettre à chacun de ses petits-enfants jusqu'à 450 000 euros en franchise totale d'impôt, tous les dix ans au lieu de tous les quinze ans, en lieu et place des 64 000 euros prévus par le droit actuel.

pourrait ainsi transmettre jusqu'à 400 000 euros en franchise totale d'impôt, qui viendraient évidemment s'ajouter aux transmissions effectuées précédemment en faveur des petits-enfants. Si c'est là votre conception des petits patrimoines, ce n'est pas celle du Gouvernement : c'est la raison pour laquelle j'ai fait part, lors des débats en commission, de l'avis particulièrement défavorable du Gouvernement sur les dispositions de cette proposition de loi. J'observe que la commission a été du même avis, parfois pour des raisons différentes, puisque, sur les dix articles que comptait le texte initial, pas moins de sept ont été supprimés. Je me réjouis que votre commission ait abandonné certaines des dispositions les plus problématiques de la proposition J'ai notamment en tête la restructuration des tarifs entre parents et enfants, qui, combinée aux élargissements des abattements proposés, pouvait conduire à alléger encore considérablement l'imposition de transmissions de patrimoines importants.

qui sont un instrument essentiel de notre politique en faveur de la gestion durable des espaces naturels. L'adoption des dispositions initiales aurait remis en cause ces outils. Si le texte issu de la commission a été allégé de la sorte, il s'est cependant enrichi, si l'on peut dire, de deux dispositions qui ne figuraient pas dans le texte initial. Ainsi, avec l'article 2, la commission des finances du Sénat propose d'instaurer une réduction de l'actif successoral à hauteur de la valeur des biens qui ont été compris dans l'actif successoral d'une récente succession ou donation dont le défunt avait lui-même bénéficié.

sur la valeur d'un bien immeuble transmis lorsqu'il est, au jour du décès, occupé par le conjoint du défunt ou par son partenaire de Pacs, ou encore par un enfant protégé du défunt. Nous ne pouvons pas davantage soutenir cette disposition : à nos yeux, le niveau actuel de l'abattement permet de tenir compte de l'impact d'une occupation de ce bien immobilier sur sa valorisation. En allant plus loin, l'on procurerait un avantage excessif, d'autant plus grand qu'il est proportionnel à la valeur du bien. Enfin, le texte issu des travaux de la commission augmente l'abattement en faveur des donations au profit des petits-enfants à 70 000 euros par petit-fils ou petite-fille, au lieu de 150 000 euros, comme le proposaient les auteurs du texte initial. Il ne modifie plus le quantum de l'exonération pour don de sommes d'argent en pleine propriété ou l'abattement général en faveur des successions ou donations en ligne directe : ce sont là autant de dispositions que nous ne pouvons approuver.

il serait d'autant moins opportun de mener ce débat maintenant que la garde des sceaux a réuni un groupe de travail interdisciplinaire appelé à se pencher sur la justification de la réserve héréditaire et sur l'adéquation de ses modalités aux évolutions juridiques et sociales. Il nous semble plus judicieux d'attendre la fin de ces travaux, qui auront un impact sur les transmissions, avant de nous lancer dans une modification de la fiscalité

L'amendement n° 13, déposé par les auteurs de la proposition de loi, vise à reprendre les dispositions de l'article 8, supprimé en commission. Il tend à mettre en oeuvre une diminution considérable de l'exonération partielle en faveur de la transmission d'entreprise, que l'on appelle parfois le « pacte Dutreil ». Il s'agit là du principal dispositif permettant d'assurer la pérennité de nos entreprises en cas de transmission à titre gratuit il vise à éviter que l'application pleine et entière des droits de mutation ne conduise à ce que les héritiers ou donataires vendent systématiquement les parts ou actions reçues, ou certaines d'entre elles, afin de payer les droits dus. Sans cela, on aboutirait à éclater l'actionnariat et la direction effective de l'entreprise, au point d'en menacer la pérennité. De surcroît, la nécessité de payer immédiatement des droits importants contraindrait les héritiers et donataires à accepter les premières offres formulées et non à privilégier la recherche de repreneurs sérieux. Ces dispositions

établissent que notre pays a connu en 2018 une hausse du taux de pauvreté, qui s'élève dorénavant à 14,7 % de la population. Selon l'Insee, cette évolution est principalement due à la forte hausse des revenus financiers des plus aisés. Ces éléments confirment clairement les récents travaux relatifs à l'impact de la suppression de l'ISF, en particulier le rapport extrêmement détaillé présenté par le président Vincent Éblé et le rapporteur général Albéric de Montgolfier. Il est désormais attesté que, sous la présidence d'Emmanuel Macron, l'on favorise les plus riches de nos concitoyens, même si M. le secrétaire d'État nous a fait grief de vouloir vouloir soutenir un peu plus certaines catégories de personnes ... Les élus du groupe socialiste et républicain du Sénat, très attachés à la cohésion sociale, s'interrogent légitimement sur cette orientation, alors qu'au cours du précédent quinquennat les inégalités avaient régressé. Les travaux de Thomas Piketty démontrent que la composante patrimoniale de ces inégalités est aujourd'hui très lourde : les inégalités sont revenues, peu ou prou, à leur niveau d'avant la Première Guerre mondiale. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une telle situation. Il s'agit d'un combat moral et républicain prioritaire, mais aussi d'un enjeu économique et social majeur. C'est dans cette perspective que notre groupe a déposé, il y a quelques mois, une proposition de loi visant à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune, et que Vincent Éblé travaille aujourd'hui à la définition d'un ISF « 2.0 », qui constituerait un outil redistributif approprié en la matière. Mais s'il est possible d'utiliser un levier fiscal au moment de la constitution du capital, il est également possible d'actionner un autre levier au moment de la transmission de ce capital d'une génération à l'autre : c'est tout l'objet de cette proposition de loi. Nous voulons adapter la fiscalité des héritages et donations afin de favoriser la redistribution. Dans cette perspective, notre texte comprenait trois enjeux. Le premier enjeu, c'est la redistribution intergénérationnelle, dans un contexte d'accroissement de la durée de vie et de recul de l'âge moyen de l'héritage en France. Patrick Kanner ayant largement développé ce point, il me paraît opportun de concentrer mon propos sur les deux autres objets. Le deuxième

Nous proposions de lisser la progressivité de l'imposition, alors que les seuils sont aujourd'hui très irréguliers. Nous proposions également, ce qui nous semblait parfaitement logique, de ne pas offrir aux mêmes héritiers plusieurs abattements dans le cas d'héritages multiples : on nous l'a également refusé. Le système actuel est pourtant aberrant : une personne qui hérite de 200 000 euros en une seule fois sera taxée au titre des droits de mutation, alors qu'une personne héritant deux fois de 100 000 euros ne le sera pas ! Comment justifier cette inégalité de traitement manifeste ? le même travail à l'article 6, afin de ne pas pénaliser les héritiers les plus modestes. Or le Gouvernement nous a opposé les difficultés de ciblage de nos propositions.

général : vous nous avez opposé le silence et le rejet pur et simple de nos propositions. Nous en prenons acte. En définitive, le deuxième enjeu de cette proposition de loi visant à assurer une fiscalité des héritages et donations plus juste et plus équilibrée a été clairement rejeté par la droite sénatoriale et par le Gouvernement. Il sera difficile d'affirmer que les plus grands patrimoines ne sont pas protégés, ce au détriment des autres parties de la population. et dernier enjeu de notre proposition de loi consistait à revoir l'assiette même des droits de mutation. Cela permettait, en premier lieu- il ne faut pas le cacher -, de financer nos propositions en faveur de la jeunesse tout en rééquilibrant la progressivité de l'impôt, et, en et, en second lieu, de mettre fin à des situations d'iniquité fiscale, voire à des pratiques d'optimisation fiscale de la part des contribuables les plus aisés. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi, aujourd'hui, l'assurance vie, premier placement financier des Français, ne serait pas incluse dans l'assiette des droits de mutation.

Comment justifiez-vous que les plus aisés puissent aujourd'hui, par le biais des placements en assurance vie, pratiquer une optimisation fiscale aussi choquante que légale ? On ne comprend pas bien non plus la subsistance du régime des bois et forêts issu de la loi Sérot, datant des années 1930 1930 : plus rien ne justifie une telle exception sur le fond. Cette niche permet principalement à quelques riches propriétaires fonciers, « agriculteurs du XVI arrondissement », de réduire leur taux d'imposition. Enfin, si nous convenons tous qu'il est nécessaire d'aider les transmissions d'entreprise familiale- je pense notamment à ce que va nous dire M. Nougein -, nous ne comprenons pas que l'on actionne le levier des droits de mutation,

mener à bien ce travail. La transmission d'entreprises, notamment familiales, peut recevoir l'appui des pouvoirs publics ; mais le système actuel ne répond pas de cette logique, et c'est cela que nous voulons changer.

de l'assiette, d'autre part ; mais nous avons trouvé un accord positif avec le rapporteur du texte, Jean Pierre Vogel, que je tiens à saluer pour le travail accompli en commission. Au-delà du débat qui a eu lieu, nous faisons oeuvre utile en favorisant la redistribution intergénérationnelle dans notre pays. Il y a lieu de s'en réjouir. Sous réserve que des amendements de séance ne viennent pas déséquilibrer le dispositif tel qu'issu des travaux de la commission des finances, nous nous abstiendrons sur la rédaction issue des travaux du Sénat : s'il est moins ambitieux que ce que nous aurions souhaité dans un monde idéal, ce texte n'en demeure pas moins une avancée utile, quoique trop déséquilibrée à notre sens, et qui ne répond pas à notre volonté originelle de plus de justice fiscale ! Très bien

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cette proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation est, semble-t-il, principalement motivée par la recherche d'une plus grande justice fiscale. Si intellectuellement on peut facilement adhérer à un tel objectif, il convient de bien évaluer les mesures proposées et d'en apprécier les conséquences économiques, sociétales et financières pour le budget de l'État.

La France a la particularité, contrairement à beaucoup de ses voisins et de pays de l'OCDE, de pratiquer une triple imposition : celle des revenus, celle du patrimoine et enfin celle qui porte sur la transmission de ce dernier. Toute modification doit prendre en compte l'ensemble des taxations, afin que les évolutions souhaitées et parfois justifiées ne débouchent pas, en définitive, sur un prélèvement global qui deviendrait confiscatoire. Il convient en même temps de ne pas priver le budget de l'État de ressources fiscales significatives dans ce domaine. C'est au nom de cette prudence et dans la recherche d'une évolution équilibrée que la commission de finances a supprimé sept des dix articles du texte initial tout en votant un article additionnel. L'un des articles supprimés concernait la réserve héréditaire ; il conduisait à diminuer la part des biens et droits successoraux dévolue aux héritiers réservataires. Cette initiative peut traduire de bonnes intentions : encourager les donations à des tiers ou mieux prendre en compte les volontés découlant de recompositions familiales de plus en plus fréquentes dans notre société. Toutefois, elle peut aussi avoir des effets négatifs pour certains types de patrimoine, dont la préservation supporte mal l'atomisation des successions. Ce sujet, qui relève autant d'une évolution sociétale que d'une question fiscale, mérite sans doute une réflexion plus large, qui était peu compatible avec une procédure de Les dispositions du texte d'origine visant à favoriser les transmissions intergénérationnelles ont bien été conservées, bien que légèrement amendées pour des raisons de rigueur budgétaire. En revanche, mesures portant sur l'intégration dans l'assiette d'éléments importants de patrimoine- parfois dans leur totalité -, comme l'assurance vie, la transmission d'entreprise ou encore les bois et forêts, ont été écartées. Sur le plan économique, ces dernières mesures semblaient mortifères pour les entreprises familiales et déstructurantes pour les biens constituant des investissements à long terme, comme la forêt. À titre d'exemple, la transmission d'une entreprise à un enfant s'accompagne souvent d'un dédommagement assuré par le bénéficiaire en faveur des autres héritiers

donc exploitables. Il convient donc de favoriser et d'alléger la charge fiscale de telles transmissions, sinon la forêt régressera dans notre pays ou deviendra essentiellement la propriété d'institutionnels et d'investisseurs étrangers.

En conclusion, la position adoptée par la commission des finances nous paraît équilibrée : préserver une ressource fiscale pour le budget de l'État sans pénaliser les donations et les successions et, au contraire, en encourageant la circulation anticipée du capital vers les jeunes générations.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est peu de dire que cette proposition de loi a suscité de vrais débats de fond au sein de la commission des finances ; mais il est vrai que l'on réveille bien des ardeurs quand il s'agit de toucher un peu au grisbi fort juste, d'un approfondissement des inégalités patrimoniales, qui viennent renforcer les inégalités de revenus- le patrimoine médian des cadres est supérieur à 200 000 euros, alors que celui des ouvriers non qualifiés s'élève à 16 400 euros nos collègues du groupe socialiste proposent de réformer la fiscalité des successions « afin de la rendre plus efficace, plus efficiente, plus juste et plus lisible ». Et il est vrai que cette question est essentielle au regard des évolutions démographiques que connaît notre pays. De nombreux économistes estiment que la réforme de la fiscalité en matière de successions et de donations sera un enjeu central des prochaines années, la question posée étant : peut-on éviter l'avènement d'une société de rentiers ? Dans le même ordre, nous ne pouvons que souscrire à l'idée d'aider la jeunesse, ou les classes moyennes et modestes ; qui serait contre de tels objectifs ? Si l'impôt sur les successions n'a pas bonne presse, comme le souligne une étude de France Stratégie citée par les auteurs de la proposition de loi et il n'en demeure pas moins que- cette même étude le souligne également -la taxation en ligne directe est largement surestimée, puisqu'elle oscille entre 3 % et 5 %, selon le montant transmis. Tout à fait. La proposition de loi initiale prévoyait, « afin de préserver le capital des ménages modestes d'augmenter de 100 000 à 150 000 euros l'abattement général existant pour les successions en ligne directe et les donations- cette mesure avait été votée en 2007 et modifiée en 2012 -, et, pour aider la jeunesse, de favoriser la transmission, que ce soit sous forme de donation ou de succession entre grands-parents et petits-enfants.

a entraîné un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros pour l'année 2008 et a représenté chaque année, à compter de 2008, près de 60 % du coût total de l'ensemble des allégements fiscaux votés depuis l'an 2000. Par ailleurs, c'est sur les notions mêmes de classe moyenne et de ménage modeste que nous sommes assez dubitatifs. Il était proposé, en effet, de soustraire à la taxation pas loin de 450 000 euros par petit-enfant- et je ne prends que cet exemple. Comme cela fut souligné en commission, si les grands-parents ont quatre petits-enfants, ce ne sont pas loin de 1,8 million d'euros qui pourraient être transmis en franchise d'impôts. Vous comprendrez que nous n'ayons pas tout à fait la même définition des classes moyennes. Comme le rappelle France Stratégie, les dispositions que vous proposez n'auraient pas d'effet sur les individus nés dans les familles n'ayant pas ou que peu de patrimoine à transmettre, qui représentent un tiers des familles. mesures n'auront d'effet que sur la moitié des individus issus de familles dotées en patrimoine. Et pourtant, ce bien eux qui composent les classes qu'on appelle « moyennes » ! Seules 12,8 % des transmissions sont d'un montant supérieur à 100 000 euros. à 100 000 euros. La revue nous rappelle que « les donations sont l'apanage des classes les plus aisées », et la note de France Stratégie enfonce le clou, ses auteurs soulignant : « Les héritages confortent les inégalités existantes au sein d'une même génération. Ainsi, les ménages ayant reçu plus de 100 000 euros d'héritage ou de donation ont des revenus courants, hors revenus du patrimoine, de 20 % à 30 % supérieurs à ceux des autres ménages.

Vous nous dites que c'est pour aider la « jeunesse de notre pays », dont l'âge de succession est de plus en plus tardif- c'est un fait. De quelle jeunesse parle-t-on lorsqu'on sait que l'héritage moyen s'élève à 67 200 euros, mais à 325 000 euros pour les 10 % les plus riches ? ? Une autre question nous semble fondamentale : pourquoi proposer une réforme qui allégerait encore considérablement la taxation de la transmission du patrimoine des plus aisés- car c'est bien de cela qu'il s'agit -au moment où l'ISF est supprimé et le prélèvement au moment, donc, où les mesures d'allégement de la fiscalité du capital n'ont jamais été aussi fortes ? Ces allégements vont coûter 4,5 milliards d'euros par an au budget de l'État, soit 22,5 milliards d'euros sur la durée du quinquennat. Et ces mesures profitent principalement à moins de 400 000 ménages parmi les plus riches, qui bénéficieront chacun d'un allégement fiscal moyen de 10 000 euros par an. C'est dans ce contexte que, sous couvert de lutter contre les inégalités intra et intergénérationnelles, il nous est proposé d'accentuer le mouvement de défiscalisation de l'héritage à l'intérieur des familles, qui a au contraire, depuis une trentaine d'années, considérablement amplifié les inégalités. Le patrimoine ne provient pas que des revenus du travail. Les revenus des capitaux contribuent à l'accumulation de richesses, surtout pour les plus grosses fortunes, celles qui sont précisément concernées par les droits de succession. Nous considérons donc que les droits de succession sont une imposition juste, qu'ils sont un facteur de rééquilibrage en faveur du travail, dans la mesure où ils permettent de réduire les inégalités de patrimoine. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait, au contraire, doter ceux qui ne disposent ni d'un capital sociologique grâce à leur entourage familial, ni d'un capital financier, d'un accompagnement de l'État sous forme d'allocation de départ dans la vie active.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je tiens évidemment moi aussi à saluer l'initiative du groupe socialiste,

Réformer la fiscalité de la succession et de la donation, c'est interroger la notion de transmission ; c'est envisager ce qu'elle implique, au niveau tant individuel que social. Le débat n'est pas nouveau ; il s'invite régulièrement au Parlement depuis la Révolution française. Mais ses termes ont changé avec le temps. L'allongement de la durée de vie, la baisse de la fécondité ou le recul de l'âge auquel on devient parent sont autant de facteurs qui soulèvent des interrogations sur la fiscalité de la transmission. Face à ces évolutions, il peut paraître utile d'adapter les dispositifs fiscaux de la succession et de la donation, mais il faut prendre garde à ne pas bouleverser les équilibres. Les facteurs que j'évoquais à l'instant s'inscrivent dans le temps long des évolutions sociétales. Le principal écueil que nous devons éviter aujourd'hui, c'est donc la tentation de nous précipiter pour tout chambouler. Sur des sujets aussi essentiels, la prégnance du problème ne justifie pas l'urgence de la solution. Elle nous appelle plutôt à la prudence. Alors que les cellules familiales évoluent, dans leur forme et dans leur structure, et alors que les parcours de vie deviennent de moins en moins linéaires, les assouplissements proposés dans la version originelle du texte pouvaient retenir notre attention et susciter le débat. Si le recul de la réserve héréditaire soulève d'importantes interrogations, d'autres aspects de cette proposition de loi pouvaient se révéler intéressants, notamment concernant l'encouragement des transmissions intergénérationnelles et la révision du barème de progressivité, autant de pistes de réflexion que nous pourrons explorer, mais certainement pas dans le cadre trop restreint d'une législation en commission. Ces pistes devraient faire l'objet d'un débat de fond en séance La fiscalité de la transmission n'est pas qu'une affaire fiscale ; c'est aussi une question sociétale. Parce qu'elle impacterait significativement le budget de l'État, parce qu'elle affecterait la façon dont les familles constituent leur patrimoine, parce qu'elle modifierait la redistribution sociale, aussi, une telle réforme devrait nécessairement se fonder sur une réflexion beaucoup plus aboutie et des travaux préparatoires plus approfondis. À défaut, je crains que nous ne confirmions, malgré nous, les craintes de ces familles qui n'y voient plus clair quant à l'avenir de leur patrimoine parce qu'elles ne comprennent plus rien aux évolutions incessantes de notre droit. Bien sûr, nul ici ne trouvera réjouissant que le travail parlementaire soit bridé par les parlementaires eux-mêmes. Que la commission ait ainsi vidé le texte de sa substance n'a donc rien de satisfaisant en soi. Mais, en tout état de cause, cette proposition de loi aura le mérite d'attirer l'attention du Parlement et du Gouvernement sur ce chantier qui se trouve devant nous. C'était manifestement, d'ailleurs, le but de ses auteurs ! Elle nous aura également permis d'affiner nos propositions et d'affirmer nos convictions. J'ai, pour ma part, et au nom du groupe Les Indépendants, suivi une ligne claire fondée sur trois principes. : réduire la pression fiscale qui pèse sur les transmissions, notamment pour les petits et moyens patrimoines, tout en assouplissant les conditions dans lesquelles les donations entre vifs peuvent être réalisées, et ce à tout âge de la vie, particulièrement entre grands-parents et petits-enfants. Deuxième principe : encourager et faciliter la transmission d'entreprise afin que nos centres de décisions et notre appareil productif demeurent en France. Il est en effet impensable de remettre en cause le dispositif du pacte Dutreil, qui est aujourd'hui la seule possibilité pour une génération de dirigeants de transmettre l'entreprise à la génération suivante, sauf, bien sûr, à vouloir en assouplir les conditions et en augmenter l'abattement dérogatoire. Il y va de l'avenir de nos PME et de nos ETI, qui structurent le tissu industriel de nos territoires. Troisième principe : avancer avec prudence lorsqu'il s'agit de modifier des dispositifs aussi importants aux yeux de nos compatriotes. Il ne suffit pas de brandir les chiffres de la répartition du patrimoine en France pour justifier l'augmentation des droits de succession ou la suppression de la réserve héréditaire. Il faut pour cela prendre le temps de mener un débat qui sera un débat de société, serein, global et approfondi, et pas seulement un débat fiscal. seulement un débat fiscal. Le groupe Les Indépendants est disposé à prendre part à ce débat, de façon active et constructive. Mais, pour l'heure, les conditions ne sont pas réunies pour prendre de telles décisions, sachant notamment que nous nous apprêtons à examiner un budget déjà placé sous le signe de la réduction d'impôts et de la maîtrise des dépenses.

que le patrimoine soit donné plus souvent- au lieu de quinze ans, nous proposons huit ans, et sans condition d'âge ; j'y reviendrai tout à l'heure lors de la discussion des amendements. Nous proposons également que la résidence principale soit exonérée à hauteur de 300 000 euros,

points négatifs, nous pensons que les allégements proposés sont insuffisants pour les petites et moyennes successions, notamment sur la résidence principale, qui est le principal bien que l'on peut transmettre, en particulier dans les familles.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'allongement de la durée de vie, dont nous devons évidemment nous réjouir, nous oblige à revoir bon nombre de dispositions. En effet, au-delà de la question de la dépendance, se pose celle de la succession. Nos concitoyens héritent de plus en plus tard. Souvent, ces héritiers sont eux-mêmes à la retraite. Je l'entends régulièrement, lors de mes déplacements : les personnes âgées sont bien souvent plus inquiètes pour leurs petits-enfants que pour leurs enfants et pour eux-mêmes.

qui propose une hausse des abattements en cas de donation ou succession entre grands-parents et petits-enfants, et même entre un légataire sans enfant et ses neveux et nièces. Car- nous ne le disons pas assez -les Français sont généreux ! Ils sont généreux lorsqu'ils savent comment est dépensé leur argent. Notons également qu'ils sont rares à faire confiance à l'État pour redistribuer les richesses.

Cela peut sembler antinomique, et ça l'est, mais, surtout, cela en dit long sur la confiance des Français s'agissant de l'utilisation de leurs deniers par l'État. L'épargne des Français atteint aujourd'hui des niveaux record, parce qu'ils n'ont plus confiance dans l'avenir. Quel nouvel impôt ? Quelle nouvelle taxe va-t-on créer ? Difficile, dans cette situation, de prendre des risques et de ne pas être dans l'expectative. Encourager les Français à transmettre leur patrimoine de leur vivant, c'est encourager ceux qui le peuvent à investir dans la jeunesse. C'est aussi, disons-le, redonner du pouvoir d'achat aux jeunes trentenaires, car, je le rappelle, l'article 2 de cette proposition de loi diminue le rappel fiscal des donations de quinze à dix ans lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 40 ans. ans. Je tiens à saluer le travail du rapporteur, mon collègue Jean Pierre Vogel, qui a su préserver les entreprises familiales, lesquelles seront d'ailleurs plus longuement évoquées par mon collègue Claude Nougein d'ici quelques instants. Cette proposition de loi est désormais équilibrée ; soulignons qu'à l'approche des discussions sur le projet de loi de finances l'équilibre est l'une des premières qualités

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, désagréable et opposé à tous mes amendements,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je souhaite évoquer l'article 8 concernant la transmission des entreprises,

Vous proposez de réduire l'abattement de 75 % à 25 % lors des successions ou donations pour les dirigeants d'entreprise qui s'engagent à garder les titres six ans actuellement. En fait, vous souhaitez voir disparaître toutes les entreprises familiales détenues par des Français, lesquelles, je vous le rappelle, représentent un emploi sur deux en France, ce qui n'est pas rien ! Tout cela, à la grande joie, j'imagine, des multinationales étrangères, qui pourront acheter à vil prix les fleurons de l'économie française. française. Si cette proposition a un impact relatif sur les TPE ou sur les petites PME, souvent faiblement valorisées, elle a en revanche un impact considérable sur les grosses PME ou ETI, les entreprises de taille intermédiaire. lors des successions, l'entreprise est valorisée par l'administration fiscale en tenant compte des plus-values latentes et non du capital investi parfois vingt ou trente ans auparavant. Malgré le taux actuel de 75 %, la France reste le mauvais élève de l'Europe en matière de transmission familiale d'ETI : 18 % seulement dans notre pays, contre 56 % en Allemagne et 70 % en Italie.

le pacte Dutreil, en gardant six ans les actions, il faut acquitter malgré tout 11 millions d'euros, ce qui est très difficile, mais pas impossible en ayant recours à des emprunts. Avec votre loi, pour la même entreprise, il y aura 34 millions d'euros de droits à payer, ce qui est impossible. La seule solution est Vous indiquez que cette vente sera une bonne chose, car « favoriser la reprise par des héritiers serait dommageable à l'activité économique ». Je rêve ! Ce n'est pas vrai : de nombreux rapports prouvent que le taux de survie à trois ans pour les transmissions familiales d'ETI est de 100 ce qui est bien supérieur aux taux de survie dans les cessions non familiales. Surtout, les transmissions familiales garantissent davantage la stabilité des effectifs. Un rapport publié en 2017 dans le cadre de la délégation aux entreprises du Sénat,

actions. J'ai vécu comme élu d'un département rural, la Corrèze, plusieurs successions d'importantes entreprises familiales qui ont dû être vendues à de grands groupes.

« au détriment des finances publiques ». Vous oubliez de prendre en compte le coût exorbitant pour les finances publiques des fermetures d'entreprises. Les coûts sociaux, économiques et fiscaux sont largement supérieurs au manque de recettes fiscales évoqué dans votre De plus, si plus tard l'entreprise est vendue, n'oubliez pas que les actionnaires paieront la plus-value. Au bout du bout, on n'échappe pas à l'impôt. Aucun cadeau n'est fait ! Enfin, l'article 8 de cette proposition de loi est à la fois inutile et nuisible.

d'instabilité fiscale et d'irresponsabilité ! Mes chers collègues, nous avons un choix crucial à faire entre prospérité économique ou idéologie fiscale égalitaire. C'est l'un ou l'autre. Il nous appartient de choisir La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. Je rappelle que les articles que les articles 3, 4, 5, 9 et 10 font l'objet d'une procédure de législation en commission. Le vote sur

À ce jour, les époux peuvent choisir le régime matrimonial de la communauté universelle en intégrant une clause d'attribution intégrale au survivant. Ils peuvent également opter pour la dotation au dernier vivant. Le conjoint survivant récupère alors la quotité disponible. Mais la part de cette quotité dépend du nombre d'enfants et peut donc être très réduite. les enfants réclament leur part au parent restant, celui-ci peut être conduit à vendre certains de ses biens- voiture ou maison. Cela entraîne de surcroît des frais notariaux nécessairement pénalisants. Dès lors que le patrimoine a été constitué par les deux parents, il n'est pas juste que les successibles puissent demander leur part avant le décès du second parent survivant. Afin de protéger ce dernier, mon amendement visait à faire de la clause au dernier vivant le principe de droit commun. Cette mesure permettait d'éviter aux parents d'aller chez le notaire et les protégeait du comportement d'enfants les contraignant à se séparer de leurs biens. Par ailleurs, seuls étaient concernés, en l'espèce, les couples mariés. Je respecte le sort qui a été réservé à mon amendement

ce qui aboutirait à un cumul d'abattement déraisonnable. À titre d'exemple, deux grands-parents pourraient donner, s'ils avaient quatre petits-enfants, jusqu'à un 1,6 million d'euros en franchise totale d'impôts tous les quinze ans. J'émets donc un avis défavorable.

M. Vincent Segouin. Le présent amendement vise à exonérer de droits de mutation dans la limite de 100 000 euros, quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur et le donataire dans les conditions suivantes : soit si les 100 000 euros sont investis à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises, à condition que le donateur exerce son activité professionnelle, au moins pendant une période de cinq ans ; soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition. Le sous-amendement n°

D'autre part, il vise à élargir considérablement le dispositif, en augmentant le montant de l'exonération de 30 000 euros à 100 000 euros et en supprimant la restriction du champ des bénéficiaires au cercle familial.

M. Vincent Segouin. En raison de l'allongement de la vie, le vieillissement de la population et conformément à l'esprit de la présente proposition de loi dont le constat et les ambitions sont justes, il semble raisonnable de supprimer l'alinéa qui dispose que le donateur soit âgé de

? L'adoption de cet amendement irait à l'encontre de l'objectif d'encourager la circulation anticipée du patrimoine vers les jeunes générations.

Aller plus loin risquerait de dénaturer le dispositif, dont l'objet consiste précisément à encourager les transmissions précoces. Après quatre-vingts ans, le donateur pourra toujours bénéficier de l'abattement de droit commun pour donner à ses petits-enfants, dont le niveau a été fortement relevé par la commission des finances.

La condition d'âge qui a été fixée, au-delà de la modification entre les soixante-cinq ans en 2007 et les quatre-vingts ans en vigueur aujourd'hui, est aussi un outil de droit pour éviter les stratégies de contournement quant aux droits de succession.

Panunzi, sur l'article. Si les quatre premiers amendements que j'ai déposés ont connu une issue satisfaisante, ce n'est pas le cas des deux derniers, qui ont été jugés irrecevables en commission. en commission. Il s'agissait en quelque sorte d'amendements d'appel visant à atteindre l'objectif de l'assainissement cadastral des territoires soumis à un désordre foncier, au premier rang desquels la Corse, territoire métropolitain le plus touché par l'indivision informelle et l'absence de titres de propriété. phénomène que l'on retrouve de façon plus marginale dans des départements tels que l'Ardèche ou la Lozère. Cette volonté d'assainissement avait débouché sur l'adoption d'une loi, votée d'ailleurs par le Sénat à l'unanimité en février 2017, dont l'article 2 prévoit que, pour les indivisions constatées dès la reconstitution du titre de propriété sur le fondement de l'article 1 de la même loi flottante, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer des actes de gestion et de conservation, qui sont titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer tout acte de disposition. Cette dérogation à la règle de l'unanimité est temporaire ; elle ne concerne que les actes établis jusqu'au 31 décembre 2027. Aussi cruciale soit-elle, elle est à ce jour inapplicable et inusitée, alors même que la période décennale est entamée de deux années. Concrètement, les professionnels du notariat ne disposent pas d'une méthodologie permettant de mettre en oeuvre cette disposition. Plusieurs sollicitations ont été adressées à la Chancellerie pour demander la publication d'une simple circulaire, en vain. Par le présent amendement, je voulais interpeller le Gouvernement, afin d'établir par voie réglementaire les modalités d'application de cet article capital pour la Corse et les autres territoires en proie au désordre foncier. J'attends donc la réponse du Gouvernement sur ce point précis. Les dispositions de l'autre amendement, qui a été jugé irrecevable, reposent sur le fait qu'il arrive souvent que les frais de reconstitution soient plus importants que la valeur vénale du bien faisant l'objet du titrement. Les frais attachés à la reconstitution des titres de propriété et aux attestations immobilières établies conformément au décret du 5 janvier 1955 concentrent plusieurs taxes dont le produit revient à l'État. La neutralisation de ces quatre taxes ne pourrait avoir qu'un impact positif en faveur de la dynamique de titrement. Sensibilisé au problème lors de son déplacement en Corse le 22 octobre 2018, et mesurant l'impérieuse nécessité d'encourager la création de titres de propriété, propriété, Bruno Le Maire a fait valoir à juste titre que lorsqu'un usager prenait l'initiative de reconstituer un titre de propriété, il devait le faire à moindre coût, voire quasi gratuitement. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement est-il prêt à s'engager en ce sens

La proposition de notre collègue portait sur une période de dix ans, avec des abattements de 10 % par an pour la succession antérieure. Je propose quant à moi un délai de trois ans, au cours duquel les héritiers pourraient bénéficier d'une réduction d'impôt.

sur l'article. Je souhaitais prendre la parole sur cet article 6 pour préciser la position de notre groupe. En effet, notre proposition de loi initiale, si elle rejoignait dans les grandes lignes l'objectif de la rédaction actuelle de l'article, était, à certains égards, plus ambitieuse. Elle permettait de protéger les héritiers les plus modestes de toute hausse éventuelle de fiscalité du fait de la modification de l'assiette et d'intégrer la donnée que représente aujourd'hui le renchérissement du prix de l'immobilier. Néanmoins, eu égard à la suppression des articles 5, 7, 8 et 9 de notre texte initial, cette rédaction, certes moins ambitieuse, nous apparaît plus appropriée pour ne pas dénaturer l'esprit de l'ensemble du texte et entraîner un effet d'aubaine généralisée. En ce sens, nous voterons l'article tel quel.

d'exonérer assez fortement la résidence principale de la succession. J'ai bien compris que l'amendement, tel qu'il est rédigé,

du Gouvernement ? Le Gouvernement partage l'avis de M. le rapporteur. J'ajoute à l'intention de M. le président Gabouty que, dans la mesure où le dispositif d'abattement proportionnel a pour objet de tenir compte d'une décote dans la valeur d'un bien immeuble à raison de son occupation,

En effet, si celui-ci a admis, en 2003, que le dispositif Dutreil n'était pas de nature à entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, c'était après avoir vérifié que « la combinaison des avantages ne peut réduire à néant les droits finalement acquittés

contre ces amendements.

Que croyez-vous que vont faire les investisseurs chinois ? Acheter les forêts françaises ! Et les troncs de hêtres, de chênes ou d'autres arbres partiront directement en Chine. Il y a une pression, actuellement, sur le marché du bois,

Les banques détiennent toujours 87 % du marché, et la concurrence ne joue pas complètement. Pourquoi ? Parce que, souvent, les assurés ne connaissent pas la date

Il s'agit de permettre concrètement au consommateur de résilier son assurance emprunteur s'il le souhaite. En effet, le consommateur apparaît souvent comme la partie faible du contrat de prêt ou d'assurance. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, depuis 2010, pour renforcer ses droits et rééquilibrer la relation qui le lie à son assureur. Plusieurs manquements sont pourtant constatés sur le terrain, qui viennent obérer les chances, pour un assuré, de changer d'assureur, donc de réaliser des économies substantielles. Mes chers collègues, avant d'examiner les solutions proposées dans le texte de notre collègue Martial Bourquin et par la commission des affaires économiques pour renforcer l'effectivité du droit de résiliation, je veux préciser de quoi l'on parle et vous donner quelques chiffres. L'assurance emprunteur est une question importante dans la vie quotidienne de nos concitoyens, puisqu'elle conditionne, dans la majorité des cas, l'obtention d'un prêt immobilier. Elle facilite donc l'accès au crédit de tous les segments de la population. Les chiffres relatifs à ce marché parlent d'eux-mêmes : 1 million de crédits immobiliers ont été contractés en 2018. À peu près autant de nouveaux contrats d'assurance emprunteur ont donc été conclus. Les cotisations de cette assurance représentent environ 9 milliards d'euros par an. En moyenne, l'assurance emprunteur représente entre 6 % et 15 % du montant du prêt pour un ménage, selon son profil de risques. Les montants en jeu sont donc considérables. Depuis 2010, le législateur est intervenu à quatre reprises afin d'ouvrir, puis d'élargir progressivement le droit à la résiliation de cette assurance, augmentant ainsi la concurrence sur ce marché. De fait, l'objectif d'une baisse des tarifs au profit du consommateur a été atteint : d'après la Direction générale ont proposé des tarifs plus bas et permis de diminuer les prix moyens, forçant les bancassureurs à s'aligner et à diminuer à leur tour les prix, afin de conserver leur clientèle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les parts de marché ont peu évolué dans les faits : si les bancassureurs détiennent toujours environ 87 % du marché, c'est avant tout parce qu'ils se sont adaptés à la concurrence, ce qui s'est traduit par plusieurs milliers d'euros d'économie pour les assurés ayant changé d'assureur. Pour autant, les intentions du législateur ne sont parfois pas respectées sur le terrain. Or il nous revient d'évaluer concrètement l'application des lois que nous adoptons et de proposer des améliorations ou des modifications lorsqu'elles sont nécessaires. En l'espèce, des incertitudes juridiques et les manoeuvres dilatoires de certains prêteurs entretiennent la confusion du consommateur, appelant des précisions et des correctifs. Une partie de ces manquements tirerait son origine du flou juridique entourant la notion de « date d'échéance » du contrat d'assurance emprunteur. Certains contrats n'en disposent pas, parce qu'ils ont été signés avant la consécration du droit à résiliation, en 2014, puis en 2017. D'autres présentent, au contraire, plusieurs dates, qui peuvent toutes en même temps prétendre à ce qualificatif. C'est ce flou qu'exploitent parfois certains prêteurs pour indiquer au consommateur qu'il n'a pas respecté la bonne date et qu'il ne peut donc pas rejoindre la concurrence. Pour répondre à ce problème, notre collègue Martial Bourquin proposait deux solutions : inscrire dans la loi de ce que recouvre la notion de date d'échéance et créer, pour les assureurs, d'une obligation annuelle d'informer l'assuré de son droit à résiliation, trois mois avant la date anniversaire de la signature du prêt. À l'unanimité de la commission des affaires économiques, des compléments et des précisions ont été apportés au texte. Je veux vous en exposer les grandes lignes. Concernant la première solution, qui consiste à inscrire dans la loi que la date d'échéance est la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur,

Par exemple, si un assuré a déjà changé d'assureur, il possède un nouveau contrat qui indique, lui, une date précise d'échéance. Il convient que l'assuré puisse opter pour cette date. La commission a donc choisi d'inscrire également dans la proposition de loi cette partie de l'avis du CCSF. Ainsi, l'assuré garde véritablement la main sur la période de résiliation qui lui convient le mieux, ce qui est un facteur de clarté et de bonne appropriation du droit

La seconde solution proposée dans le texte consistait à créer, pour les assureurs, une obligation d'informer l'assuré trois mois avant la date d'échéance de son droit à résiliation. Bien informer le consommateur est fondamental, car c'est seulement ainsi que celui-ci connaîtra ses droits et pourra faire jouer la concurrence. Toutefois, nous nous sommes rendu compte que, présentée ainsi, cette obligation ne pouvait tous les assureurs ne connaissant pas cette date de signature de l'offre de prêt, qui relève des relations contractuelles entre un prêteur et un emprunteur. Ainsi, pour les contrats en cours, qui sont parfois anciens, les assureurs seraient contraints de calculer une période d'envoi de l'information à partir d'une date qui leur est inconnue.

pour la bonne information du consommateur. C'est pourquoi la commission a choisi de créer une obligation pour l'assureur d'informer chaque année l'assuré de son droit général à résiliation et des délais et procédures qu'il doit respecter s'il souhaite en faire usage. Ainsi, chaque assuré saura qu'il peut résilier son contrat et sera informé de la démarche à accomplir, à charge pour lui, bien évidemment, de connaître sa date de signature. C'est un vrai pas en avant dans le rééquilibrage des relations entre le consommateur et l'assureur. Il a également été décidé de renforcer fortement les sanctions administratives dans les cas où les prêteurs et assureurs tentent d'induire leurs clients en erreur, de ne pas leur répondre ou de le faire hors délai, bref, de les tromper de mauvaise foi. En effet, une obligation sans sanction risque de rester un voeu pieux, à l'opposé de ce que nous recherchons. Aujourd'hui, les sanctions pénales s'élèvent à 3 000 euros environ. Non seulement leur montant est trop faible, mais elles sont peu appliquées dans la pratique. La commission les a dépénalisées, afin que la DGCCRF et l'Autorité soient en charge de les appliquer. Cela présentera un avantage décisif : leur montant s'élèvera jusqu'à 15 000 euros par infraction pour une personne morale, soit cinq fois plus qu'aujourd'hui. En outre, le droit actuel offre à la DGCCRF et à l'ACPR la possibilité de publier leurs décisions de sanction, pour plus de dissuasion. Voilà, mes chers collègues, le travail conduit par la commission des affaires économiques. Je me félicite que ses propositions aient été adoptées

le crédit immobilier est un élément essentiel de l'accès à la propriété de nos concitoyens. Il est, à ce titre, un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. Plus de 9 millions de ménages disposent aujourd'hui d'un crédit immobilier, pour un encours cumulé de plus de 1 000 milliards d'euros, à des taux historiquement bas. Dans ce contexte, la capacité pour nos concitoyens à trouver une assurance pour leur prêt immobilier qui les protège à un coût acceptable est évidemment importante. C'est la raison pour laquelle le législateur s'est très légitimement intéressé aux modalités de souscription des contrats d'assurance emprunteur depuis plusieurs années. Les réformes qui se sont succédé depuis 2010 ont permis des avancées significatives. La loi du 1 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a introduit une évolution importante, avec le principe de la déliaison déliaison entre le prêt immobilier et l'assurance emprunteur, sous réserve que la garantie soit d'un niveau équivalent. Ce dispositif a ensuite été renforcé par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, qui a renforcé les droits du candidat à l'assurance emprunteur, pour garantir sa liberté de choix, par la loi du 17 mars 2014, qui a octroyé à l'assuré la possibilité de changer d'assurance emprunteur à tout moment jusqu'à douze mois après la signature de l'offre de prêt, enfin, par la loi du 21 février 2017, qui a ouvert la possibilité de résilier un contrat d'assurance emprunteur chaque année pendant toute la durée du prêt. Grâce à ce cadre législatif très étoffé, les emprunteurs peuvent désormais choisir l'assureur de leur choix et substituer une nouvelle assurance à l'assurance initiale selon une périodicité annuelle. La loi prévoit également une information renforcée des emprunteurs qui leur permette d'éclairer leur décision. La remise systématique d'une fiche standardisée d'information, la FSI, et la création du taux annuel effectif de l'assurance, le TAEA, facilitent la comparaison des offres. Le Gouvernement est attentif à l'effectivité de ces réformes, qui sont attendues par nos concitoyens. La possibilité de déliaison et de substitution d'assurance emprunteur a permis une modération des primes d'assurance pratiquées et réduit la charge financière pour les emprunteurs. Dans l'avis qu'il a rendu le 18 avril 2017, le Comité consultatif du secteur financier a confirmé que ces évolutions avaient permis d'accroître la concurrence sur les marchés. Toutefois, des difficultés sont apparues dans la mise en oeuvre du droit de résiliation annuel du contrat d'assurance. En effet, les contrats groupe d'assurance emprunteur signés avant le 1janvier 2018 ne comportent pas de date d'échéance annuelle. Or cette date fait courir un délai de deux mois au cours duquel l'emprunteur peut demander, chaque année, la résiliation de son contrat. En l'absence de date d'échéance, il n'est pas possible aujourd'hui aux emprunteurs concernés d'exercer, dans les faits, leur droit à la substitution. Nous avons confié au Comité consultatif du secteur financier la mission d'identifier une solution à cette difficulté pratique. Je salue l'excellent travail de cette instance, qui réunit des représentants des professionnels de la banque et de l'assurance, des associations de consommateurs, des parlementaires et les pouvoirs publics, pour arriver à des solutions

Le comité a ainsi retenu la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur, sauf en cas de demande d'une autre date par le client, si celle-ci existe contractuellement. L'accord obtenu en 2018 formalise également l'engagement des assureurs d'étendre la durée des contrats d'assurance jusqu'à cinq ans en cas d'allongement de la durée du prêt. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez souhaité, avec cette proposition de loi, inscrire dans la loi l'accord auquel le CCSF est parvenu sur la date de résiliation annuelle, mais aussi renforcer les modalités d'information de nos concitoyens et clarifier le régime de sanctions applicables, pour assurer une effectivité sans faille de ces réformes.

Si, aujourd'hui, les taux de crédits immobiliers sont historiquement bas, avec 1,25 % en moyenne hors assurance, les prix d'achat sont de plus en plus élevés. Cette situation amène les ménages à emprunter beaucoup d'argent. La Banque de France, d'ailleurs, s'en inquiète. Le taux d'effort des ménages a connu une augmentation importante ces dernières années, avec un peu plus de 30 % des revenus consacrés, en moyenne, au remboursement des échéances.

extrêmement importante pour de nombreux ménages qui se sont engagés ou qui vont s'engager dans un prêt immobilier pour quinze, vingt, voire vingt-cinq ans. Je ne reviens pas sur les propos tenus par notre collègue Martial Bourquin, que je remercie de sa ténacité. Il nous a rappelé l'histoire législative des dix dernières années sur le sujet.

Ce gain peut donc être très important quand on sait que l'endettement des ménages français bat des records. La négociation de l'assurance emprunteur doit permettre un véritable gain de pouvoir d'achat pour les emprunteurs. Elle est même souvent la variable d'ajustement pour réussir à boucler un plan de financement dans un contexte où l'accession à la propriété

qui aide les jeunes ménages à acquérir leur premier logement. La suppression du PTZ sera vécue comme une nouvelle injustice pour les familles qui vivent dans les zones périurbaines et dans nos campagnes. J'en reviens à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Oui, les marges sur les assurances emprunteur sont énormes. Oui, ce marché reste capté par les banques. Un tiers des ménages ont un prêt immobilier en cours et 80 % d'entre eux disposent d'une assurance souscrite auprès de leur banque. Nous arrivons à un point de bascule, le coût de l'assurance emprunteur devenant plus élevé que celui du crédit lui-même. Par exemple, pour un crédit de 250 000 euros sur vingt ans, de quarante ans versera 35 000 euros d'intérêts, mais 36 000 euros pour l'assurance emprunteur. Or le marché de l'assurance emprunteur rapporte près de 9 milliards d'euros, compte tenu de la dynamique des prix de l'immobilier. L'encours total des prêts liés à l'habitat a, en effet, franchi le seuil symbolique de 1 000 milliards d'euros en fin d'année dernière. Depuis dix ans, pour tenter d'ouvrir ce secteur à la concurrence et faire baisser les prix. Dès lors, pourquoi le secteur ne s'ouvre-t-il pas à la concurrence ? Pourquoi proposons-nous de légiférer encore ? Il faut que

embrouillés, à l'avenir, sur la date de résiliation de leur contrat. Ce point devrait faire consensus, Mme le rapporteur ayant proposé de reprendre la liste que le CCSF avait négociée avec les banques, les assureurs et les associations de consommateurs. En outre, l'information du consommateur sera renforcée. Tout d'abord, la date de résiliation sera précisée dans la notice que le prêteur est obligé de fournir à l'assuré au moment des premières simulations. L'emprunteur aura connaissance de ses droits dès le début du processus de souscription d'un prêt. Ensuite, et c'est là un point essentiel, nous créons une obligation annuelle d'information du client sur son droit à résiliation et les modalités d'exercice de ce droit.

s'il souhaite engager une démarche de renégociation de son contrat. Sur proposition de Mme le rapporteur, l'article 2 met en place un régime de sanctions administratives plus efficace, voire dissuasif : la DGCCRF pourra appliquer des amendes allant jusqu'à 15 000 euros par manquement constaté, soit cinq fois plus que l'amende actuelle. Ce qui est très important également, la DGCCRF aura la possibilité de rendre publiques ces sanctions, le fameux qui fait souvent plus peur aux entreprises que les amendes. Enfin, je tiens à rappeler que les mesures adoptées ont vocation à s'appliquer aux contrats en cours.

Il est utile de clarifier la notion de date d'échéance en entérinant dans la loi l'avis du comité consultatif du secteur financier, le CCSF. L'obligation de faire apparaître cette date dans la notice annexée au contrat de prêt constitue une avancée pour les contrats nouvellement conclus. Outre les confusions autour de la date de référence pour l'exercice du droit de résiliation, les associations de consommateurs constatent la persistance de manoeuvres dilatoires visant à décourager l'emprunteur. décourager l'emprunteur. Il s'agit notamment du non-respect, par les établissements de crédit, des délais de réponse quant au refus ou à l'acceptation du nouveau contrat, de la non-précision des documents manquants et de l'absence de véritable motivation du refus de changement.

apporte des explications, critère par critère, sur l'absence d'équivalence des garanties entre le contrat de groupe et le contrat individuel. Le contenu de l'information annuelle de l'assuré a été complété en commission par les modalités de résiliation du contrat et les délais à respecter. Toutefois, tel qu'il est rédigé, rédigé, l'article concerné ne permet plus de savoir à quel moment doit intervenir cette information. Je crains qu'elle ne soit délivrée trop tardivement. Or cette précision est essentielle, puisque le rapport dispose que les délais de résiliation peuvent s'élever jusqu'à Nous avons donc déposé un amendement visant à ce que le délai de trois mois, retenu par la proposition de loi initiale, soit applicable aux contrats nouvellement conclus. L'assurance emprunteur a toujours relevé d'un droit particulier pour ce qui est des conditions de résiliation. Presque dix ans après la reconnaissance du droit à la déliaison, nous sommes encore en train de légiférer sur le droit à la résiliation, nous rapprochant un peu plus du droit commun. Faudra-t-il aller jusqu'à un alignement sur ce dernier, à savoir la résiliation à tout moment sans justification ? Certes, il conviendra ultérieurement d'évaluer les effets de la déliaison sur la mutualisation des risques, donc impact sur les profils à risque, qui intéressent moins les assureurs. Pour l'instant, la démutualisation n'a pas entraîné d'augmentation des contributions de ces catégories. La demande de rapport est ici pertinente.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la présente proposition de loi s'inscrit dans la lignée des différentes réformes du marché de l'assurance emprunteur initiée par nos collègues voilà maintenant plus de dix ans. Elle vise à parachever cet effort, en clarifiant et en renforçant l'information du consommateur sur son droit à la résiliation. L'assurance emprunteur est un véritable enjeu, au coeur de la vie de nos concitoyens. Elle représente une part importante du coût de leur crédit, souvent conditionnée à l'obtention du prêt immobilier. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises ces dernières années en ouvrant, puis en élargissant progressivement le droit à la résiliation, augmentant ainsi la concurrence de l'offre. Le constat est aujourd'hui simple : le manque d'information du consommateur persiste. Il existe un réel besoin de clarifier la date retenue lorsqu'un assuré souhaite faire usage de son droit de résiliation. La date anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur apparaît alors opportune. Aussi, je félicite le travail de la commission, qui a jugé utile d'offrir au consommateur la possibilité de choisir une autre date, afin de garder la main sur la période de résiliation qui lui convienne le mieux.

tout au long du crédit. Elle est particulièrement utile au consommateur pour connaître les exigences minimales du prêteur et, ainsi, comparer les offres d'assurance. nous voterons l'amendement du Gouvernement qui tend à supprimer la disposition imposant au prêteur de communiquer, sur demande de l'emprunteur, la fiche standardisée d'information. Cette disposition est en effet déjà satisfaite par le code de la consommation pour les cas de substitution avant l'offre de prêt. Enfin, le texte propose de créer pour l'assureur une obligation annuelle d'informer l'assuré sur le droit général à résiliation et sur les modalités de mise en oeuvre. Obliger l'assureur à informer le consommateur trois mois avant la date d'échéance, comme cela était proposé initialement, aurait été une contrainte trop importante pour les assureurs qui ne connaissent généralement pas cette date. Mes chers collègues, ces mesures de bon sens vont permettre une bien meilleure information du consommateur. Ne pas être entravé lorsqu'on souhaite faire usage de son droit à résiliation est une question non seulement d'égalité et de légalité, mais surtout de pouvoir d'achat. Cette réforme était nécessaire. Je tiens à remercier le travail fourni par Martial Bourquin, Élisabeth Lamure et les membres de la commission. Les échanges fructueux nous ont permis de partager de manière unanime l'objectif de ce texte. Ainsi, le consommateur pourra réellement faire jouer la concurrence. La concentration des acteurs du marché de l'assurance emprunteur reste toujours problématique et porte aujourd'hui préjudice aux consommateurs en termes de pouvoir d'achat.

Madame la présidente, madame la secrétaire

Les assureurs se sont parfois montrés réticents à laisser leurs clients partir vers la concurrence. Certains font traîner en longueur le traitement des demandes de résiliation ; d'autres jouent sur la complexité et sur l'obscurité des dispositions contractuelles. Leur but est de dissuader ou de gêner les consommateurs dans l'exercice de leur droit de résiliation. Même en l'absence de telles manoeuvres, les consommateurs sont encore trop souvent dans l'ignorance de leurs droits. Mal informés ou gênés dans leur volonté de changement, ils restent trop souvent liés à la banque qui leur a accordé un prêt et fait souscrire une assurance. Cela explique sans doute pourquoi cette activité d'assurance de prêt, qui pourrait être effectuée par n'importe quel assureur, est aujourd'hui encore très majoritairement l'apanage des prêteurs bancaires. La libre concurrence est un principe auquel le groupe Les Indépendants est très attaché. Elle permet aux consommateurs d'exercer leur liberté de choix en même temps qu'elle garantit des prix raisonnables. C'est en partie le cas dans le domaine des assurances de prêts. Les prix ont déjà commencé à baisser, mais il subsiste une importante marge de progression. L'étape incontournable vers davantage de concurrence est l'information du consommateur quant à sa faculté de choix. Les dispositions du texte la renforcent utilement. Les obligations sans sanction n'obligent personne. C'est presque aussi vrai des sanctions dérisoires. Nous nous réjouissons donc que la commission ait quintuplé les sanctions encourues. Portées à 15 000 euros par infraction, elles devraient avoir les propriétés dissuasives que nous leur souhaitons. Fallait-il dépénaliser les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ? Nous comprenons bien que ce passage d'une sanction pénale à une sanction administrative vise l'efficacité. Et nous ne doutons pas de la compétence de la DGCCRF, ni de celle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, dans la mise en oeuvre de contrôles et de sanctions, même si déléguer des fonctions de justice à l'administration L'ensemble du texte est équilibré et nous semble correspondre aux attentes du secteur. L'économie de marché, le libéralisme économique ne signifient pas l'absence de règles. Ils ont au contraire besoin de régulation, d'encadrement et de contrôle. Sans cela, la concurrence peut rapidement tourner à l'abus de position dominante ou au cartel. C'est par le droit que nous pouvons nous assurer que la concurrence demeure loyale, que les acteurs bénéficient de la meilleure information et que chacun respecte les règles du jeu.

sans doute d'achever la réforme de l'assurance emprunteur entamée en 2010 par la loi Lagarde et complétée, quatre années plus tard, par la loi Hamon. Les ambitions de ces réformes et de cette proposition de loi sont cohérentes et constantes

Aujourd'hui, le changement d'assurance emprunteur est encore insuffisamment utilisé, et la concurrence ne joue pas à plein. La situation s'est améliorée, mais elle reste variable d'un profil d'emprunteur à l'autre. Nous devons être vigilants pour que les possibilités de changement ne bénéficient pas qu'à un public sans risque et nous montrer garants de l'équité entre chacun. Ainsi, le renforcement des obligations des assurances et des banques en matière d'information du consommateur sur ses droits à résiliation est le bienvenu. Mme le rapporteur des modifications apportées qui nous rassurent sur la faisabilité concrète de cette réforme. Le flou sur la date d'échéance est dissipé : le texte permet à l'assuré de la fixer lui-même.

l'assurance représente toujours entre 6 % et 15 % du coût du crédit. Cette proportion est loin d'être négligeable. Nous constatons même qu'elle augmente avec la baisse historique des taux d'intérêt il devient parfois plus coûteux de s'assurer que d'emprunter. Ce rapport entre les deux coûts liés à un crédit nous interroge. Nous devons mettre en garde les prêteurs de ne pas profiter de taux d'intérêt bas pour augmenter le coût des assurances. Finalement, le consommateur pourrait sembler gagnant sur le montant total, mais le prêteur assureur ne ferait pas complètement jouer la concurrence. La protection

Je souhaiterais ainsi nous mettre en garde collectivement contre certaines dérives de notre système. La recherche du coût le plus bas possible ne doit pas se faire au détriment du niveau et de la qualité de l'assurance. En outre, nous devons faire attention à ne pas renchérir le coût des assurances emprunteurs sous prétexte de nouvelles contraintes pour les assureurs. ces derniers ne peuvent prétendre à une charge sur une mission qu'ils ont mal assurée jusque-là. Enfin, madame la secrétaire

Comme souvent, le contrôle nécessite des moyens budgétaires et humains. Nous examinerons bientôt le projet de loi de finances pour 2020. Et même si nous vous faisons confiance, nous observerons avec attention les moyens qui seront mis à disposition.

mon ancienneté au Sénat me permet de garder un souvenir assez net des avancées à la fois progressives et poussives dans le domaine de l'assurance des prêts. Il a tout de même fallu cinq lois pour que cette chasse gardée des banques rentre enfin dans le droit commun de la résiliation des contrats d'assurance La loi Lagarde, en 2010, a pour la première fois inscrit la possibilité de souscrire une assurance de prêt dans l'établissement de son choix. Mais il a fallu tout de suite que la loi Lefèvre précise que le choix d'une assurance en dehors de la banque prêteuse ne pouvait causer de frais additionnels pour l'emprunteur. En 2015, la loi Hamon fut, selon moi, à la fois une percée et un échec. Elle ouvrait timidement la voie de la résiliation, mais seulement dans le court délai de douze mois suivant la signature d'une offre de prêt, alors que ladite loi rendait complètement libre la résiliation des assurances auto et habitation, pourtant bien moins lourdes pour le consommateur. Deux ans après, le Sénat se rebiffe et introduit dans la loi Sapin le droit de résiliation que le Conseil constitutionnel invalidera après saisine des banques, soucieuses de ne pas perdre leur pactole. Mais notre collègue Bourquin n'abandonne pas et fait voter un amendement qui va enfin permettre la résiliation annuelle, y compris pour les contrats anciens. Ce sont des milliers d'euros que vont ainsi pouvoir économiser les emprunteurs immobiliers, s'ils font l'effort de réaliser une mise en concurrence réelle.

En effet, les banques elles-mêmes proposent maintenant des taux comparables à ceux des assureurs alternatifs. L'ouverture à la concurrence a eu cet effet bénéfique.

Vous l'avez compris, j'applaudis ce texte qui devrait constituer, je l'espère, la dernière étape de ce long parcours que je suis depuis presque dix ans. Si j'interviens, c'est aussi pour exprimer mes convictions et mes réserves. améliorer l'information des consommateurs emprunteurs doit être une préoccupation constante du législateur. Mais, dans une économie très concurrentielle, où tous les coups sont permis, nous ne devons pas non plus nous comporter comme des nounous.

depuis le 1 janvier 2018, les emprunteurs peuvent résilier l'assurance décès de leur crédit immobilier pour faire jouer la concurrence et diminuer les coûts. Plus d'un an après, le résultat espéré n'est pas à la hauteur. Après analyse du marché, on s'aperçoit que les banques ont usé de tous les moyens possibles pour dissuader leurs clients de partir. Seul un public averti y a eu recours. Les moyens employés par ces mêmes banques n'ont d'ailleurs pas tous été loyaux ... Nous ne

emprunteurs. Dès 2017, la fédération des banques s'est opposée en contestant, auprès du Conseil constitutionnel, la validité des mesures adoptées par la loi. Elle a aussi combattu les recommandations sur les bonnes pratiques à adopter fixées par l'ACPR. Ces démarches ont été infructueuses, mais elles auront permis aux banques de gagner du temps pour organiser la défense de leur portefeuille. Assez vite, par le jeu de la concurrence, les clients ont compris qu'ils avaient souscrit un contrat groupe collectif avec un taux unique, quel que soit l'âge des souscripteurs, alors qu'ils pouvaient avoir un contrat individuel fondé sur l'âge des souscripteurs et sur leur situation. Le contrat collectif est donc très lucratif pour les banques. Nous comprenons pourquoi ces dernières ont craint l'ouverture du marché. Pour décourager les clients, mais aussi la concurrence, elles ont utilisé différentes méthodes : contestation de la date de résiliation, absence de réponse aux résiliations,

Cette disposition est indispensable pour éviter à l'avenir les litiges et contentieux sur les résiliations. Sur l'article 2, j'ai émis de fortes réserves, considérant qu'il était compliqué pour l'assureur d'adresser un courrier spécifiant la date d'échéance, le délai et les modalités considérant, aussi, que c'était contraire au bon fonctionnement d'une société commerciale. De fait, la mise en place de ces documents d'information va contraindre l'assureur à revenir chaque année sur le contrat, à renégocier les conditions et à augmenter ses frais de gestion, ce qui peut faire perdre une partie du bénéfice de la réduction des coûts attendue par les emprunteurs.

à l'article 3- le fameux ... Autant je comprends la motivation de notre collègue Martial Bourquin, déçu par les résultats de la loi et les moyens employés pour la remettre en cause, autant je suis rassuré que le rapporteur ait supprimé cet article.

? Une décision tacite d'acceptation emporte des conséquences potentiellement très lourdes. Certes, le prêteur qui ne répond pas dans les dix jours manque à son obligation, et ce manquement doit être sanctionné par la DGCCRF ; mais une décision tacite d'acceptation par le prêteur n'est pas souhaitable, car elle pourrait créer des situations dans lesquelles un prêt

la présentation distincte dans l'offre du remboursement du prêt et de l'assurance. Quel est l'avis de la commission ? Dans tous les cas, une négociation technique sur la substitution de contrats d'assurance a lieu entre l'assureur délégué choisi par l'emprunteur et le prêteur. Ce sont des négociations entre professionnels. Ce qui compte réellement, pour que le consommateur ne soit pas captif de sa banque, c'est sa bonne information sur son droit de changer d'assureur. Or cette information est aujourd'hui correctement communiquée aux consommateurs et elle le sera davantage encore si la proposition de loi

ne sont plus à démontrer. Je propose donc d'obliger les assureurs à présenter l'intégralité des motifs de refus dans leur décision initiale.

répond à des pratiques constatées par les associations de consommateurs. Lorsque la demande de résiliation est refusée par l'établissement de crédit en raison de documents manquants, ces derniers doivent être explicitement mentionnés. De même, si le contrat alternatif est refusé au motif de l'absence d'un niveau équivalent de garanties, l'assuré doit pouvoir obtenir de la banque une véritable motivation du refus du contrat d'assurance alternatif.

En revanche, il est vrai que certaines décisions de refus sont prises au motif que des documents manqueraient dans la demande de délégation formulée par le consommateur, sans qu'il soit précisé de quels documents il s'agit.

Si l'information de la banque intervient un mois avant la date d'échéance, il sera déjà trop tard : le contrat repartira pour une année, privant l'assuré de l'effectivité de son droit. La date d'échéance des anciens contrats étant, semble-t-il, méconnue, cette mesure s'appliquerait aux contrats nouvellement conclus après l'entrée en vigueur de la loi.

au plus tôt et au plus tard trois avant la date choisie par l'assuré. Ainsi, cette information ne risquera pas de tomber dans les oubliettes de sa mémoire.

en commission, adopté à l'unanimité. Elle permettra de renforcer efficacement l'information du consommateur, sans créer une obligation trop complexe pour l'assureur, qui

l'article 1 de la proposition de loi prévoit que la date d'échéance est, au choix de l'assuré lorsqu'il souhaite résilier, la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt ou une autre date si elle figure sur son contrat.

Cet amendement tend à supprimer la demande de remise d'un rapport au Parlement évaluant, d'autre part, l'impact de la réforme de l'assurance emprunteur depuis la loi de 2014 relative à la consommation, dite part, le fonctionnement de ce marché, ainsi que son degré de concurrence. Le Comité consultatif du secteur financier, le CCSF, réalise régulièrement des bilans et émet des avis sur l'assurance emprunteur. Il a déjà dressé un premier bilan sur l'équivalence du niveau de garanties en assurance emprunteur en avril 2017, qui nous a d'ailleurs permis de travailler sur ce texte. Il a d'ores et déjà prévu un nouveau bilan en 2020. Cette instance réunit des représentants du Parlement, des professionnels du secteur financier, des représentants du personnel et des représentants des clientèles du secteur financier, ainsi que des personnalités qualifiées, notamment des universitaires.

Par ailleurs, la loi contraint le CCSF à transmettre son rapport au Parlement. Dans ces conditions, je pense qu'il faut éviter les doublons. Aussi, la commission a émis un avis de sagesse.

loi a été adoptée à l'unanimité des présents. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique a été publiée. Cette candidature sera ratifiée